dans la discussion des articles. Nous sommes parvenus à l'amendement numéro 159 au sein de l'article 2. Et une série de d'explication de vote était engagé qui se sont interrompues à la coupure que nous allons reprendre et je passe tout de suite la parole à notre collègue Cécile Cukierman. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord. Précisé et bien évidemment nous ne voterons pas Monsieur le Ministre, cette suppression de l'article de pour le dire avec beaucoup d'élégance, c'est un petit peu supprimer cet article de la proposition de loi déposée ce serait comme supprimer l'article 7 de la loi dont nous avions débattu la semaine dernière elle perd tout son sens et je crois que les débats qu'il y a eu notamment avant. La coupure donne à voir effectivement la vision en tout cas qui est proposé, à travers cette proposition de loi, est-ce que finalement on est dans une logique certes qui vise à assembler un certain nombre de collectivités, avec une vision assez descendante ou est-ce qu'au contraire on construit de par la réalité des territoires communaux. Les besoins et donc les différents arbitrages. Je ne veux pas bien évidemment ici rouvrir les débats que nous avons eu. Au moment de la loi notre au moment de la fusion des régions mais cela a été dit précédemment, avant la coupure. Oui, aujourd'hui nous avons 13 grandes régions avec des compétences renforcées et et je veux rappeler que contrairement à ce que certains ont dit avant la coupure. La décentralisation, ce n'est pas organisé une reconcentration territoriale. Et et soyons voilà faisons dit très attention collectivement. Parce que à vouloir à un moment donné à voir des, des régions qui deviennent des super-. Régions qui décide de tout et qui impose finalement aux élus locaux dans leur territoire un aménagement du du territoire on créera d'autres soucis, d'autres difficultés, et en l'état, nous ne voterons pas cet amendement. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, pour vous dire que nous non plus nous ne vendrons pas cet amendement néanmoins quelques. Quelques précisions. Je pense qu'il ne faut pas qu'on caricature non plus la la réalité locale. Il s'avère que encore ici dans cette salle, il y a des élus régionaux ou des élus qui l'ont été il pensé qu'il ne représente pas non plus les territoires. Je pense que c'est un, un peu simple. Deuxièmement, le problème de nos régions. C'est pas tant. La situation qui est celle qui est la leur. Actuellement, c'est le fait que nos régions quand on les compare à ce qui existe dans le reste de l'Europe sont à la fois impuissante et sans moyens et c'est notre c'est la vraie difficulté et que si un jour on veut qu'il y ait un pouvoir fortement décentralisé en France forcément les régions en feront partie, et on devrait s'en réjouir. Mais la vraie difficulté, Monsieur le Ministre, c'est que ici votre principe via. Contrevenir à un des principes essentiels d'une certaine façon de la décentralisation et qui est tout simple, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les collectivités territoriales françaises et d'une certaine façon. Avec votre proposition vous instaurer une hiérarchie de la région vers les autres niveaux, alors même que nous pensons de manière je pense transpartisane est majoritaire que c'est bien. Par la négociation que la région pourra jouer son rôle pleinement et non pas dans une logique verticale qui fait que d'une certaine façon les territoires. Considéré alors comme le ben subalterne n'auraient plus leur mot à dire et en ce sens. Il nous semble que cette proposition est mauvaise. C'est pour ça que que nous ne la voterons pas pour rester à l'équilibre qui a été trouvé par le texte qui nous est proposé ce soir, je vous remercie. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, moi j'écoute ces débats avec intérêt. Élu de de. L'Île-de-France et donc d'un territoire très urbain. J'avoue que je n'ai pas nécessairement l'appréciation qu'ont mes collègues. Sur d'autres territoires et d'autres régions. Mais je voudrais faire 2 remarques, d'abord je comprends les demandes de plus d'autonomie du bloc communal et notamment de la commune lorsque j'étais maire d'Arcueil. J'ai parfois rêvé de déclarer la république autonome d'Arcueil. Les textes ne m'ont pas permis de le faire et peut-être était-ce plus sage parce que dans la crise climatique que nous vivons. Si j'ai une certitude, c'est que nos destins sont liés et qu'il a absolument nécessité d'un travail itératif entre l'échelon régional l'échelon national aussi d'ailleurs dans tous les cas entre l'échelon régional et l'échelon communal sur les sujets qui qui nous occupe et moi c'est ce que je voudrais défendre ici dans, dans notre hémicycle c'est que ce dialogue devrait être la règle. Alors évidemment la création des très grandes régions a sans doute beaucoup affaibli. En en rompant des Liens historiques et géographiques et et c'est comme ça, peut être que je traduis les réticences que j'entends. Sur les bancs de la majorité sénatoriale. Mais il n'empêche que, chers collègues. Nos destins sont liés et qu'on ne peut pas sur les sujets. De biodiversité eau d'alimentation. Réfléchir dans un Isola communal non plus donc sans doute il y a dans la définition des modes et des procédures de dialogue la nécessité d'apporter des réponses qui rassurent le bloc communal et qui garde une cohérence et une convergence à l'échelle régionale qui n'est pas une échelle jacobine mais plutôt une échelle girondine que personnellement j'appelle de mes voeux. Non, non. Monsieur Folliot. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre. La loi train a été une catastrophe hein pour les territoires. Au niveau de la République. Ça a été une catastrophe pour les régions, notamment pour celles qui ont été. Obligatoirement fusionner et moi je prendrai l'exemple de la région Occitanie qui est très vaste, et puis pour laquelle il n'y a plus aujourd'hui. Ce ce ce ce lien qui était déjà. Assez disparates avant la région Midi-Pyrénées était déjà la plus grande de France paraît. Les l'étendue géographique et avec la région Occitanie, si vous me permettez l'expression, c'est pire. Ça c'est le 1er point le 2ème point. Ça a été une catastrophe aussi en obligeant la fusion de l'intercommunalité. Pour avoir des territoires qui ne correspondent plus à des éléments de bassin de vie quotidienne et et de proximité avec tout ce que cela représente somme toute avec votre proposition. Monsieur le Ministre vous allez remettre si vous me permettez l'expression, une pièce dans la monnaie. Ou dans le monde en fait donner un petit peu plus de légitimité, surtout sur une compétence qui n'est pas la sienne parce que plusieurs collègues lundi et l'ont rappelé fort justement tous les éléments relatifs à à l'urbanisme à l'habitat. Ce sont des compétences qui sont dans le bloc communal et que donc dans ce cadre-là, il eut été plus sage. De confier cela à l'échelon intercommunal départemental. Ah. A minima, peut être. Mais je crois que nous sommes face à un cadre qui assurément n'est pas sage. Il est temps de le corriger et donc c'est pour cela que la proposition qui est faite. Par madame la présidente et monsieur le rapporteur. Au niveau de la Commission spéciale au travers. De de de de de leur proposition me paraît plus sage et plus pertinente pour nos territoires. Merci monsieur le rapporteur. Parce qu'on a terminé avec les explications de vote, des collègues. Oui, monsieur le président. En fait si on en est là, c'est-à-dire à demander une prise en compte et non pas une mise en compatibilité c'est que les régions n'ont pas vraiment différencier non pas vraiment de territorialiser non pas vraiment discuter des demandes de propositions. Faites par les Scott. Et finalement on en est à se dire que. Accepter la compatibilité c'est accepter la planification. Alors certes si entre temps les régions du Yémen, chef de file de la transition écologique. Bien sûr, mais accepter ce fascicule réglementaire avec une mise en compatibilité c'est accepter une machine qui va devenir de plus en plus folles, c'est-à-dire des sera être contraignant qui vont gérer l'urbanisme alors que je n'ai pas la compétence de la région qui vont gérer le logement. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire, De plus en plus de compétences avec la biodiversité à son terme. Alors pourquoi pas. Entre temps, on a un décret qui va intervenir le premier. Les premiers ont posé problème. On verra bien le prochain sur la nomenclature donc hein sera d'être contraignant un décret sur la nomenclature une digitalisation de l'appréciation de l'artificialisation

et puis au bout un règlement européen. Une directive européenne, ça va se passer au mois de juin pour. Aller plus loin sur le sujet de la la biodiversité et la protection des sols. Je m'attendais pas sur ça c'est pas tout à fait le débat de ce soir. Mais si on accepte le schéma planificateur avec son fascicule réglementaires. Il faut se mettre en compatibilité c'est accepter cette histoire qui va se poursuivent comme ça donc. Le Sénat est bel et bien le dernier endroit où on va parler encore de confiance dans les élus de liberté locales. Mais c'est pas une façon de sortir Dusan c'est une façon de dire. À travers la prise en compte fait confiance aux élus, on s'inscrire par eux-mêmes dans les trajectoires. Il y a des rendez-vous il y a un contrôle de légalité, qu'on se rassure, les les élus seront au rendez-vous de l'histoire. Ils sont dans la sobriété foncière déjà. Voilà donc sous ses sous ses mots la prise en compte ou mise en compatibilité se joue toute cette histoire là aussi. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Au commencement était la Convention citoyenne et la Convention citoyenne a dit on va prendre la maille communal. On va prendre chaque commune et on va diviser par 2. Sa trajectoire. Les parlementaires dans le cadre de la loi climat et résilience ont dit non parce que la moitié de zéro, ça fait 0, parce que ceux qui ont fait des efforts vont pas. Pouvoir être récompensé. Donc il faut qu'on différencie et con territorialisée et le choix qui a été fait, ça a pas été de donner ça l'État mais à des élus. De faire confiance à des élus et le choix qui a été posée à ce moment-là, ça a été de confier cette responsabilité au conseil régionaux. Je me retrouve dans la situation un peu baroque. De défendre des majorités régionales qui ne sont pas toutes nécessairement les plus proches du gouvernement sur le plan de leur composition dont vous préjugés par anticipation qu'elles ne tiendront pas compte de la réalité locale. Dont acte. Ce que je dis c'est que après avoir voté l'article 1 qui dit, il faut laisser davantage de temps à la concertation. Je considère que précisément le fait de laisser à la maille régionale cette responsabilité avec du temps permettent d'avancer. Il y a trois niveaux théoriques dans un sera dettes. Il y a la prise en compte. Il y a la compatibilité et il y a la conformité. Le choix fait. Pour vous c'est d'aller vers la prise en compte pour nous, c'est pas d'aller vers la conformité qui serait une forme de tutelle c'est d'aller vers la compatibilité et l'aménagement du territoire qui a été abondamment évoqués est une compétence régionale pas l'urbanisme mais l'aménagement du territoire et si on remonte le temps avant dettes il y avait les directives territoriales d'aménagement. C'était l'état qui, par décret en Conseil d'État fixait les trajectoires. Je pense que ce serait pas un progrès en termes de décentralisation de revenir vers ce schéma. Ce que je dis c'est que en vous assurant d'un délai vous vous êtes assuré des moyens d'avoir une discussion. Et que si on passe de la compatibilité à la prise en compte, c'est l'effectivité du dispositif que nous menaçons ce qui nous pose une difficulté parce que la biodiversité peut pas attendre et que autant nous avons à faire en sorte de veiller à ce que ce soit intelligent et souples dans l'application. Autant si on va sur ce niveau de souplesse à ce moment-là, c'est plus de la souplesse, c'est du détricotage de l'assurance de pouvoir tenir les objectifs et les ambitions. J'entends que ça n'est pas la position majoritaire mais la franchise c'est de vous dire à haute voix à la fois ce que je pense, et ce qui me semble être le point majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, quand la commission mixte arrivera je respecte évidemment la légitimité totale de la haute assemblée de défendre le bloc communal. Je dis que si on avait trouvé le schéma qui permettait d'aller négocier directement avec les communes, ça se saurait. Parce qu'on a de telles différences de trajectoire entre celles qui gagnent de la population et celles qui en perdent, celles qui ont des friches et celles qui n'en ont pas qu'une maille supra communal a fini par devenir un point de consensus et explique qu'on en soit arrivé là. Ce que je souhaite c'est qu'on reste à ce point du texte, climat et résilience, je pense que ça donne du poids et de la cohérence à ce qui a été votée et ce qui va l'être. Merci. J'ai encore une demande d'explication de vote Madame Lienemann. Ministre que vous visez l'efficacité par votre méthode plaidant sur l'idée que celle proposée par le Sénat ne le serait pas. je vais vous dire, je pense exactement l'inverse. Et c'est une longue expérience d'élu local. Confronté à des nombreux schémas à l'époque c'était les Sdrif d'eau je crois essentiel. Que le document de base partent d'une volonté communale. Qui se confronte donc on en prise en compte en dialogue. Avec les instances régionales. Puisque c'est la région le sujet. Je ne crois absolument pas à l'obligation de compatibilité ou de. Pourquoi, parce que quand vous avez un document qui ne vous convient pas que vous êtes dans une commune. Qu'est-ce que ça produit. D'abord du blocage. Et jamais dû faire. 80% de nos grands document contraignant. Ont amené des blocages. en rien modifié stratégiquement les pratiques. Je me rappelle. La région Île-de-France. Les documents régionaux devait nous protéger contre l'urbanisation doigt de gant vous savez le long des mon oeil ça a rien protégé du tout. En revanche ça empêcher un développement plus harmonieux de certains secteurs qui aurait pu le faire. En clair sur ce dossier là, il me semble que si on veut que Lausanne deviennent progressivement une pratique, efficace et partagée. Il faut que ça parte d'un dialogue de basse entre les collectivités locales, notamment les communes et les régions et que ce soit l'obligation si je puis dire, d'une forme de consensus jamais totalement consensuel mais de large accord qui prévalent car sinon on construira plus de logements on sera bloqué dans du développement économique et on aura de toute façon pas réellement réaliser les objectifs de biodiversité. Donc moi je soutiens pleinement la proposition initiale de notre commission du Sénat et je crois, Monsieur le Ministre merci la tentation technocratique prévaut trop souvent dans ce genre de document. je vais prendre un exemple pour essayer de vous convaincre du bien-fondé de la strate régional. Elle ne Valérie Létard va me comprendre lorsqu'on nous a annoncé dans les Hauts-de-France, que le canal Seine Nord arriver les agglomérations se sont regroupés ensemble dans un organisme, une espèce de Pôle métropolitain des agglomérations du Nord Pas de Calais qui était basé sur le neuf, neuf Birmanie. Et parce que. On voyait dans les territoires qui avaient la compétence de logements économique. Il y avait des centaines de friches industrielles en bord à Canal on s'est rendu compte que si on se mettait pas autour d'une table et et de dire attention à ce qu'on fait le canal Seine Nord va arriver chaque territoire va essayer de récupérer de son intérêt personnel. Un petit bout de quelques hectares avoir Canal pour faire du développement économique et en en termes très vite brader les terrains et donc, cette organisation qu'on avait mis en place au 9 9 bis. On a fait un, un bilan de toutes de tous les terrains économiques encore à Canal et ensuite qu'est-ce qu'on a fait on l'a donnée au conseil régional en disant c'est à vous qu'il avait la compétence des le mois économique de hiérarchiser les priorités de développement économique en bois Canal faisons confiance un organisme intermédiaire qui la région parce que d'abord ce sont des élus ou on nous y avons-nous représentant précisément de voir au mieux possible. C'est cette problématique que l'on discute ce soir. Hein. Merci Monsieur Salmon. Merci monsieur le président, chers collègues. Des élus, il y en a sur toutes les strates effectivement le maire est un élu de de proximité. Mais c'est un élu qui est un homme comme les autres qui n'est pas infaillible, qui est soumis à des pressions qui a aussi des faiblesses. De devoir répondre à un certain nombre de d'injonctions contradictoires et on on le sait bien, les maires parfois ont des égo qui le leur, qui les ont amenés à faire une salle d'une salle des fêtes. Alors qu'il y en avait une autre dans la commune à côté on l'a vu pendant des piscines, enfin bon, si tout cela n'est pas infaillible, on a des objectifs qui sont devant nous. On peut se dire que chacun va jouer sa partition et qu'à la fin on aura une belle symphonie mais personne n'en est sûr. Quand on a plein de quand il y a pas de chef d'orchestre, il y a quand même des difficultés et je pense que la région même si j'entends bien tout ce qui a été dit tout à l'heure, on a des régions qui ont été. Qui ont été. Et qui ne correspondent plus, aujourd'hui à des territoires. Reconnus par les habitants et cela pose des problèmes bien entendu mais il y a un moment je pense qu'il faut y ait quelque chose de prescriptif, sinon on va se retrouver, hé bien avec. Chaque mère qui va faire au mieux chez lui mais est-ce qu'on va atteindre des objectifs. Je ne le crois pas. Donc c'est pour ça que moi je je je plaide pour avoir un véritable chef d'orchestre d'et la région, à mon avis, est le plus pertinent. Bien merci. Donc je pense qu'on va pouvoir passer au au vote après toutes ces explications de vote. Donc je mets aux voix. L'amendement 159 amendement de suppression présentés par le gouvernement, avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour. Cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient. N'est pas adopté. Nous passons l'amendement 188 présenté par Monsieur Dantec. Oui mais, merci Monsieur. Monsieur le Président. Donc un amendement qui va dans le même sens, mais qui renforce quand même. Les éléments de dialogue. C'est un peu la différence avec l'amendement qu'a présenté Monsieur le Ministre, qui était un peu. Excusez-moi monsieur le ministère peu brutal dont la suppression de de l'article qui est de maintenir notamment le fait que la région doit justifier par écrit ses choix. Par rapport notamment à tout l'amont. Autour de la conférence Interscope tout ou un terrain than je crois que c'est, c'est important effectivement qu'on soit extrêmement attentif à ce qui se passe en amont parce que c'est là que ça se, ça se joue donc il faut renforcer la concertation il fallait, il faut aller sur un projet partagé pour que derrière effectivement. Ce. Ce sera, dette. Puisse être accepté et déclinée dans les territoires avec la compatibilité qui n'est pas la conformité parce que je trouve que certaines des interventions ressemblent plus à un refus de la conformité qu'un refus de la compatibilité parce que les tribunaux administratifs sont extrêmement souple

Plus généralement, je trouve qu'on a un débat extrêmement intéressant. Je crois qu'il y a un quasi consensus du Sénat pour détricoter les régions telles que Manuel Valls les a proposé ce qui n'était pas l'idée initiale de la loi notre ne l'oublions pas. Marylise Lebranchu avait une autre vision quant à la lancer cette réforme que les méga-régions que Manuel Valls nous a imposé donc en tout cas il y a un consensus ici pour redécouper la France, c'est déjà une grosse avancée de ce débat et nous serons extrêmement intéressé par vos propositions et ensuite je crois que quand on voit l'évolution de la France. Et quand on voit l'évolution de l'Europe, pour reprendre le le sens de l'histoire de Jean-Baptiste Leblanc a bien décrit, c'est quand même les endroits où les régions sont fortes en termes d'aménagement du territoire et de planification qui s'en sortent le mieux aujourd'hui mais ça nécessite d'où le sens de cet amendement un travail étroit avec les autres strates. Avis de monsieur le rapporteur. Pour la commission. La. Monsieur le président, il s'agit du même amendement de suppression que le précédent, donc ce sera défavorable. Merci Monsieur le Ministre. Sagesse parce que fondamentalement, on aura un sujet avec cet article 2, le moment venu donc donner le sentiment qu'on est capable de le réécrire alors qu'on a une ligne de front potentiel sur le caractère prescriptif ou non prescriptif me pose une difficulté pour l'enrichir. Donc un avis défavorable de la commission un avis de sagesse du gouvernement. Y a-t-il des demandes d'explications de vote non, je n'en vois pas. Donc, je le soumets aux voix qui est pour l'article 188. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté 2 amendements identiques en discussion commune. Le 7 rectifié bis. Il est présenté par Monsieur Blanc.

Dans votre proposition. Et vous revenez sur les dispositions du décret du 29 avril. Et qui prévoit que les prescriptions en matière de Nona de non-artificialisation. Seront inscrites dans le sera Dans. Les rapports d'objectifs et non plus dans les fascicules comme le prévoyait le décret. Et on voit bien ici qu'il existe une opposition. Entre celles et ceux qui souhaitent que. Ces schémas soit extrêmement prescriptif et rentre dans le détail, ce sont les tenants de l'inscription dans les fascicules et puis celles et ceux qui pensent que les régions doivent avoir une certaine liberté qu'elles doivent poser des principes et ensuite avec les collectivités de base se mettre d'accord. Et en fait on va opposer. Ces 2 thèses. D'un côté on veut être précis et de l'autre côté, on veut plus de liberté Les régions ne sont pas les mêmes. Dans celle-ci, il faut peut être être extrêmement prescriptif parce qu'il y a une pression folle sur les territoires. Dans telle autre, les choses sont peut être complètement différente. Pourquoi ne pas accepter cette diversité. Pourquoi ne pas accepter que les régions que les conseils régionaux choisissent l'inscription dans telle ou telle les dispositifs du sera dette c'est une liberté Quelle décentralisation veut on veut une décentralisation qui fait confiance aux régions. Où veut-on une décentralisation qui est une fausse décentralisation qui leur impose qui les contrôle. tout cela sous le contrôle du juge administratif. Alors l'amendement que j'ai déposé. Il est inspiré par les régions de France. Il vous propose une chose pour une fois en matière de décentralisation, de faire confiance à la liberté.

De ce qui est le, la meilleure formule mais au stade du débat et après la déclaration du ministre qui dit, tout cela est est un peu tôt, je le retire pour justement éviter toute ambiguïté dans le débat ce stade. Bien, donc il ne reste que l'amendement de secte cette rectifié bis monsieur le rapporteur. Quel est votre avis. Monsieur le Président, j'ai longtemps partager le point de vue d'Étienne Blanc qui je n'ai aucun lien de famille et je le reprécise pour la millième fois.

et la prise en compte. Laisser à la carte, c'est une option qu'on avait étudié. Mais que nous n'avons pas retenu. Au final, cette commission spéciale donc en l'état. On maintient notre position de de se battre pour une prise en compte et on demandera un retrait ou sinon ce sera un avis défavorable. Monsieur le Ministre. Le paradoxe, c'est que je partage tellement l'intervention d'Étienne Blanc que j'étais pour faire confiance aux régions leur laissant la responsabilité de prescription et donc on se retrouve avec un front renversé avec un Jean-Baptiste Leblanc qui ne soutient pas votre amendement parce que ça reviendrait à se rapprocher de la position du gouvernement et moi qui ne peut pas le soutenir parce que c'est moins 10 ans que la position du gouvernement mais peut-être qu'il y a quelques pistes dans votre amendement pour faire en sorte de rapprocher demain. Députés et sénateurs autour d'une position régions de France serait entendu.

Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés.

bien que je sois contre le principe je suis toujours attachée à ce que ce soit mieux rédigé même quand c'est défavorable. Donc c'est pour ça que je transforme mon défavorable en sagesse. Si ces rédactions. Donc un avis de sagesse du gouvernement. Donc il est pour l'amendement 250. Qui est contre. Qui s'abstient il être adopté je mets aux voix l'article 2. Qui est pour. Qui est contre. Olivier. Qui s'abstient. Il est adopté. Donc amendement après l'article 2, le 114 rectifié. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, de la Corse est un document majeur d'aménagement du territoire. Cependant. À ce stade de la procédure de révision reste lourde et sape l'agilité nécessaire à un aménagement durable et vertueux. À ce jour en l'absence de procédure de révision simplifiée du Padduc telle qu'elle existe pour les plus reste fastidieuses. Et voire dissuasive empêchant cet outil d'atteindre sa pleine potentialités. C'est pourquoi le présent amendement entend permettre une procédure de révision simplifiée dans un nombre de cas limités définis par l'Assemblée de Corse. J'ajouterais par ailleurs qu'une telle procédure permettrait d'intégrer les diverses évolutions législatives relatives à l'urbanisme afin de mettre en conformité plus rapidement les documents d'urbanisme des communes. Et des intercommunalités ou encore des plans régionaux. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président et chers collègues, alors il nous semble que la loi climat résidence permet déjà d'employer la procédure de révision du Padduc maintenant plus légère et plus et plus lorsqu'il s'agit d'intégrer Elsa donc sur le principe je comprends néanmoins votre souhait que la Corse plus bénéficier de procédures encore plus. Accélérer. Cependant, il nous semble aussi que la votre amendement défini le Champ auxquels ces procédures dérogatoires pourrait s'appliquer ni le détail de ces. Procédures puisque c'est renvoyé des délibérations de l'Assemblée de Corse. Lors de l'examen qui la loi climat résilience nous avons refusé que les régions déterminent elles-mêmes les procédures de modification du sera tête pour intégrer Lausanne nous avons inscrit ces procédures dans la loi, donc on prend des, j'en suis sûr que nous ne pouvons pas faire mettre une aussi large dérogations au seul bénéfice de la collectivité. De Corse même si nous l'aimons beaucoup. Donc ce sera un avis de retrait ou défavorables. compte tenu du fait que ça n'est pas précisément relié à l'objet Dusan il y a déjà une procédure de modification allégé qui existe sur Pau aussi sur possibilité de l'Assemblée de Corse et donc pour les mêmes raisons. Ma position est la même sur ce certains sur cet amendement que le rapporteur demande de retrait sinon défavorable. Monsieur par Engie retrait donc. Donc, l'amendement est retiré. Nous passons à l'article 3 avec l'amendement 61 rectifié bis monsieur Billac. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre. Voilà la présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Donc cet amendement a pour objet. De. Supprimer cet article. Qui concerne donc. La conférence régionale de gouvernance. Parce que je pense qu'on a déjà. Suffisamment d'Erstein. Et que là on va créer dans chaque région. Le conférence du le le territoire avait 50ème membres plus par département. Chez nous on a 13 départements. J'ai vu dans les amendements. Pourquoi pas, qu'on ajoute déjà des représentants des offices HLM. Pourquoi pas des représentants de l'argent pour la culture, bref comme disait le général de Gaulle, on va créer un marché Qui vont se réunir avec un cabinet qui préparera le document. Je ne pas il ne veut pas que les maires euros donc j'attends beaucoup parlé depuis le début de la fois réussir. Soit pas même d'obtenir quoi que ce soit de cette instance. Et donc nous avons déjà.

Moi il me semble que depuis qu'on parle de simplification. C'est de plus en plus compliqué. Et c'est plus un millefeuille. Ah c'est un million de feuilles territorial, que nous avons. s'il vous plaît, n'en rajoutons pas. Je pense que nous en avons assez pas caution demander à nos concitoyens, ceux qui page toutes les instances. Je pas ce que nous dirait que c'est beaucoup d'argent des impôts pour rien. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le président. Chers collègues leur. Évidemment, ce sera un avis défavorable mais juste un mot ou est-ce que vous êtes.

À la commission des finances pour le financement Dusan qui est un sujet tout aussi important, évoqué la possibilité d'une agence Dusan voilà dès qu'on prononce certains mots ça ne, ça ne va plus, donc voilà c'est. Donc c'est un peu facile d'écarter comme ça parce qu'il y a un vrai besoin. Et quel est ce besoin. c'est de mettre les élus autour de la table. Voilà, on ne peut pas laisser l'État seul décider de qu'est-ce qu'un projet d'intérêt national, qu'est-ce qu'un projet d'intérêt régional la gouvernance au au quotidien de Dusan nous semble qu'il est pas mauvais d'avoir des élus autour de la table pour représenter toutes les catégories d'élus mais il me semble aussi que c'est pas forcément inutile. Le bloc communal. Le Bloc intercommunal le bloc départemental et y compris ceux qui ne sont pas dans ce, dans des documents d'urbanisme, donc je suis maire rural voire très rurales voire hyper rural je ne suis pas dans son document d'urbanisme voir j'ai du mal à me faire entendre demande Interco une alité de mon Scott et encore plus de ma région. Ben c'est une façon de défendre une position à travers la conférence régionale avec des représentants des élus. Alors après, qu'il faille calibré. Bien pensé. Améliorer. Sans aucun doute. Nous ne pensons vraiment enfin. Collègues pourront peut-être vous contredire mais que dans cette commission spéciale. C'est une idée forte qui s'est dégagée que de mettre en place une gouvernance Dusan voilà pour y mettre de ben non seulement des élus, mais de la souplesse en se donnant rendez-vous en appréciant des trajectoires. En mettant. De la souplesse. On reviendra sur cette souplesse plus tard peut-être. Donc c'est pour ça que je maintiens un avis. Parce. Très défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Les handicaps dont vous les affubler que se tienne ses conférences régionales. Je pourrai savourer le fait que justement après avoir expliqué que il y avait trop de normes on rajoute une instance. Et on va passer un certain temps à discuter de qui doit en faire partie, qui ne doit pas en faire partie jusqu'à combien il avait qu'un nombre qui sera le même. Globalement, quelle que soit à la fin, la taille des régions leur périmètre. Et avec les mêmes arguments que vous entendrez de ceux qui n'en font pas partie en considérant que c'est pas représentatif parce que tous les territoires non pas une voix au chapitre. Et qu'on a en quelque sorte confisquées à une partie d'échelle régionale le débat. Mais l'autre côté, j'entends que si nous n'avons pas une structure de concertation. Qui permet d'assurer un lien et on ne pourra pas le faire, entre tous les maires du territoire et la région. On a sans doute un chaînon ou un maillon qui peut manquer dans le fait de pouvoir y compris suivre l'application du dispositif. Donc. Je vais me réfugier dans la sagesse. Considérant que vous avez souhaité. Qu'on crée un dispositif qui fassent davantage d'aller retour. Vous proposer un dispositif qui est cohérent avec la manière dont vous venez de réécrire l'article de mais qui va soulever sur toute une partie du territoire. Les objections qu'ont été faites et qui amèneront. Là où vous avez mis une souplesse, une forme de complexité, c'est un équilibre qui se comprend donc je comprends la cohérence de la position du rapporteur et de la commission. En restant dans la mienne je ne peux pas ne pas vous faire part de ses doutes pour vous expliquer la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à ce projet. Bien merci donc je vais soumettre monsieur Billac. Oui, mes chers collègues. Moi j'entends monsieur le rapporteur. Mais nous n'avons de dénoncé les lourdeurs administratives. L'inflation normative toutes les contraintes qui pèsent ici ou là. Et là où nous avons le pouvoir de décider. Nous créons une conférence si la fait Genève ne remplit pas son rôle, on le supprime la faire l'je crois et ont créé un compte rage régional mais ne rajoutons pas ne rajoutons pas ne rajoutons pas c'est de l'argent public ou ça mes chers collègues. Bien merci. Je vais soumettre cet amendement on voit. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons à quatre amendements identiques en discussion commune. Le 160 rue 168 rectifié pardon madame Nathalie Delattre. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent amendement propose de maintenir dans chaque région. La conférence les conférences des Scott actuel qui ont tout de même bien fonctionné comme le rappelle le rapport de la commission spéciale pour mémoire. Elles sont composées de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale des structures chargées de l'élaboration des schémas de cohérence territoriale siège également dans cette conférence de représentants des EPCI et des communes compétentes en matière de documents d'urbanisme et non couverts par un Scott. Pour rappel, l'article 194 de la loi climat et résilience prévoit d'ores et déjà qu'elles établissent un bilan de l'intégration et de la mise en oeuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation nette au plus tard trois ans après leur dernière réunion. Plutôt que de déstabiliser l'existant. Le présent amendement propose de répondre aux critiques relatives au manque de transparence et Alain fut suffisante, association des autres communes et intercommunalités. Il propose ainsi la mise en place de groupes de travail composés de maires et présidents d'artère communalité intéressé représentant la diversité des territoires. Il établit par ailleurs un lien entre les travaux des conférences régionales des Scott au niveau régional et ceux des commissions de conciliation des documents d'hormones d'urbanisme au niveau départemental. Grâce à l'association des représentants des collectivités siégeant dans ces dernières, je vous remercie. Merci madame la présidente. Un autre amendement présenté par Madame Espagnac l'171. Oui, monsieur le président, c'est il s'agit du même amendement donc que Madame Delattre qui vise donc à

Et il est défendu très fortement par l'Association des maires de France. Donc il faudra en tenir compte. Merci et donc il n'y a plus que trois amendements parce que le quatrième il y a pas de signataires présent pour le défendre mais ils sont identiques. Allez-y monsieur le rapporteur. monsieur le président, alors. Merci à tous les collègues qui porte le message de l'AMF. C'est évidemment une option qu'on a étudié. Les les conférences Scott ont souvent fait un excellent travail ça gêne nullement de le remettre en cause. À telle enseigne que c'est ici au Sénat qu'on a choisi les squats comme l'échelon le plus pertinent. Donc surtout qu'on se rassure sur l'océan, le sort des Scott. Voilà. Il s'agit simplement de savoir si on associe les élus ou pas. Alors est-ce qu'on les associe par la voix de groupes de travail moi ce qu'on les associe formellement dans une conférence régionale, la commission spéciale a tranché parce qu'il nous a semblé que c'est un message qui est

des avis à la région et puis ce sera simplement des avis et nous en reparlerons aussi. Et puis puisque on est sur le sujet pour pas alourdir le débat je vais devancer aussi des amendements à venir auquel je proposerai un avis favorable qui laisseront. La région les EPCI et les communes déterminer ensemble la composition de leur conférence régionale. Sur un modèle qui existe déjà. À propos des intercommunalités un accord local et la loi. Peut-être qu'on pourrait laisser mais je vais laisser notre collègue nos collègues de développer un petit peu plus tard. Donc voilà. Conférence et Scott des élus. Et puis une liberté qu'on va essayer de d'instiller dans ce dispositif, qui soit une réussite. Donc en l'état ce sera demande de retrait ou défavorables. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Sagesse. Sagesse de Monsieur le Ministre, Monsieur Lemoine. Merci beaucoup monsieur le président. On voit bien que l'amendement proposé par par nos collègues à l'instant. S'inscrit dans la même dynamique que celle qui était la commission celui d'associer les élus. Et qu'il est, il peut il peut peuvent tout à fait cohabiter avec le le texte de l'article 3 de la commission. Puisqu'il s'agit d'impliquer encore plus d'élus. Il s'agit Isère impliqué à travers des groupes de travail parce que la, que la conférence se réunissent effectivement quatre, cinq, six fois pour faire des propositions, c'est une chose mais c'est encore plus intéressant, me semble-t-il de faire vivre cela. De façon plus élargie. C'est ce que propose. Ces amendements de façon assez transpartisane. Le texte de la commission peut s'en trouver utilement enrichi. Sans que ça nuise au dispositif qui a été adopté en commission. Oui, monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Réunir les maires dans une X ième conférence moi je comprends très bien mais mais quel pouvoir vont-ils avoir parce que il y a une chose qui arrive de plus en plus souvent, c'est de la réunionite, sans aucun pouvoir effectif sur les décisions qui vont être prises, c'est-à-dire que est-ce que cette conférence va pouvoir. Influer sur les décisions qui sont prises sur les permis qui sont refusés sur les périmètres et cetera parce que si c'est encore de la consultation sans aucun résultat. Je crois que les maires et notamment dans les territoires ruraux. On a vraiment assez ce type de de parodie qui semble leur donner du pouvoir et en fait ne leur donne

Oui, merci Monsieur le Président, sur l'Monsieur le Ministre je juste pour. Être certain d'avoir bien compris que si si un de ces amendements. Est adopté, ils font tomber tous les autres. On est bien d'accord, donc je voulais juste attirer la l'attention de de de tous mes collègues que. Même si on on a on a un intérêt particulier pour le travail qui est réalisé dans la conférence des des on vote cet amendement on crée. Un pouvoir délibératif à la conférence Scott qui aura, lui, demain le la responsabilité de pouvoir. Donner des des directives sur sur les territoires aux communes ou aux uns, aux intercommunalités moi je crois à la légitimité de l'élu à la légèreté démocratique, on peut contester le choix de la région ou pas de la région aujourd'hui le sera être il est fait par la région, il y a une instance qui a été. Proposé par le par le texte et par le rapporteur qui est sous la responsabilité de l'instance qui met en oeuvre le sera dette c'est-à-dire la région. Je voudrais juste attirer votre attention. Sur sur le fait que si ces amendements sont sont en fait a priori tomber tout le reste et on confie. À des gens qui n'ont pas forcément la légitimité démocratique. Le choix de faire des des de prendre des orientations très importantes pour l'aménagement de notre territoire. Oui. Moi je je voterai cet amendement qui me semble assez au-delà du débat compatibilité aux prises en compte. Je crois qu'on est. Assez d'accord globalement enfin de ce que j'ai compris des débats pour dire qu'en amont. Du document. Du sera il faut quand même qu'on discute beaucoup plus avec l'ensemble des élus et des strates concernés, c'est-à-dire y compris créer une culture régionale de l'aménagement qui ne peut pas être le seul fait des élus régionaux. Donc je trouve cet amendement va tout à fait dans ce sens-là et je le je le voterai. Je ne pense pas qu'il fasse tomber un amendement sur le nom derrière de la. De de cette commission. Mais je pense que la, la, la commission spéciale a fait oeuvre utile en créant quand même un lieu de travail et je crois que l'idée d'groupe de travail ça approfondit quand même donc c'est pas juste un bidule qui se réuni. Pour finaliser un document. Ça veut dire qu'il y a un travail approfondi de cohérence à l'échelle de la région avec des des gens qui ont qui ont une vraie expérience de terrain et que en termes démocratiques on va tout à fait dans le bon sens, ça veut dire aussi derrière que la région puisque on a entendu des critiques fortes sur la technostructure des des méga- régions finalement d'une technostructure qui soit dégagé de la réalité des élus locaux, c'est ce qu'on a entendu. Avant la pause. Je crois que si on a une commission représentative. Au contraire, on ne pourra pas avoir un document régional d'aménagement derrière qui soient dégagé du travail de cette commission, vu la composition qui est proposée. Donc je crois que ça va tout à fait dans le bon sens. Et après il aura le débat compatibilité o prise en compte. Donc je crois que effectivement de ce côté-là, je crois que la commission spéciale est en train de créer un mécanisme qui compris participera peut-être d'une vision régionale partager plus forte par rapport aux critiques qui ont pu s'exprimer. Tout à l'heure. je voulais dire que je je je j'entends bien ce qui se dit sur cette conférence régionale des Scott qui a d'ailleurs joué parfaitement son rôle, enfin dans les territoires où elle a pris la peine d'être transparente et de, de réfléchir. Avec avec tous tous tous les Scott et les EPCI non couverts. Sur ces questions, mais quand on parle de l'échelon régional de la loi, on ne parle pas de la collectivité, région cet échelon régional ça défense stratégique et encore une fois le. Le réfléchir à cette échelle-là c'est pas complètement incohérent avec le fait de pas donner tous les pleins pouvoirs au conseil régional pour décider à la place de toutes les collectivités qui. Qui sont à l'échelon inférieur en outre dans la conférence régionale des Scott. Il y a pas le il y a pas les départements et on voit bien les conseils départementaux ont quand même toute une place à jouer, ils sont en charge. De l'équité territoriale de la solidarité territoriale et et très clairement on a besoin d'avoir leur parole aussi présente et puissante pour traiter de cette question du zéro artificialisation nette donc la conférence régionale de Scott A. a son rôle à jouer mais pour avoir une, une et, une bonne échelle et est une bonne instance de 10 libération de choix. De choix d'avenir, de choix d'arbitrage de soit de répartition de choix des grands projets de choix des petits projets de là où on consomme ou pas l'enveloppe, hé bien je pense que cette conférence est bien plus compétente que la conférence régionale des Scott.

La proposition qui est faite toutefois néanmoins est cependant, je pense que s'il y a possibilité de considérer que la conférence des Scott peut être un lieu de débat et de véritables concertations. Moi j'ai tendance à préférer l'idée du concept d'accord local qui est très souvent des pendus, défendue par le Sénat éperonné qui permet au niveau à l'échelle d'un territoire régional et non pas décrété par la région de pouvoir organiser la conférence régionale des Scott de manière la plus pertinent j'aurais un amendement tout à l'heure qu'il est le 10. Rectifier terre qui permet à la fois de satisfaire la demande qui est formulée là mais qui permet surtout de prendre en compte la diversité des territoires et la libre administration des territoires. Donc pour ma part je ne suis pas favorable à ces amendements qui pourrait être je pense largement satisfait par celui que je vais présenter qui est encore plus large et plus souple. Merci monsieur le président, chers collègues. Peut être aussi. Ajouter que. À ce stade-ci. La commission spéciale a souhaité travailler sur une conférence régionale Dusan associant les élus et les différentes strates d'élus territoriaux. C'est aussi, Monsieur le Ministre, parce que dans la volonté. Qui s'est exprimée par le décret d'application mis en oeuvre par l'administration centrale. Nous avons changé le sera d'être de nature. Un changement total de paradigme. C'est devenu un schéma prescriptif qui va s'imposer à tous les documents d'urbanisme et comment voulez-vous que face à cela, les associations d'élus. L'ensemble des intervenants que nous avons pu entendre n'aient pas souhaité pouvoir être associé. Une instance de dialogue qui va arbitrer. Décider de ce qui va s'imposer dans leurs propres documents d'urbanisme et donc je pense que c'est la suite logique des discussions et de l'état de l'ARC a reçu effectivement le Parlement suite aux évolutions qui ont été mises en oeuvre dans les décrets, donc effectivement cette traduction dans la gouvernance Dusan cette association des élus à leurs sous une forme qui est un peu plus. on va dire direct que la proposition de maintenir une conférence des Scott avec des groupes de travail, c'est que dans des groupes de travail, les élus locaux. On va pas leur demander d'exprimer un avis le seul la seule entité qui resteraient en lien Direct avec les régions. Ce sont les Scott. Les élus, les représentants des collectivités n'aurait pas ce lien Direct. C'est pour ça qu'il nous semblait que. À ce stade il n'était pas souhaitable et l'Association des maires de France n'ailleurs ne s'oppose pas à la proposition de gouvernance Dusan du tout et nous pensons que l'amendement que Françoise Gatel propose apportera des souplesses un dispositif général qui est celui que nous avons initiée collégialement dans notre texte de la commission spéciale avec une possibilité effectivement de faire valoir un choix différent s'est partagé de façon consensuelle et large avec les collectivités. donc avant de passer aux amendements qui vont suivre et 11 amendement on va d'abord voter sur les trois qui seront proposées là le 168 le 171. Et le 200 avec un avis donc défavorable de la commission un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés. Donc on passe maintenant la discussion. Commune sur les 11 amendements qui suivent le 1er présenté par Monsieur Vial 76 rectifié. Oui, merci Monsieur le Président c'est c'est effectivement un amendement de de souplesse que que je vous propose, puisque il reprend quasiment telle quelle la la composition de de la conférence. Dusan que souhaite la Commission. En ne précisant pas en revanche le nombre de représentants par catégorie. Tout simplement parce qu'effectivement les régions ne se ressemblent pas. Qu'. En Bretagne par exemple, j'ai appris récemment que toutes les communes étaient couvertes par un Scott et donc il n'y avait pas forcément de sens de rendre obligatoire la présence d'une commune représentant un territoire qui n'étaient pas couverts par un Scott. On a des territoires très large comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, que je connais bien avec des territoires de montagne qui nécessitent ne reprend activité spécifique des la métropole de Lyon, qui elle aussi à une des des spécificités et donc l'objectif c'est de laisser à la région. qui présidera cette conférence comme le vol texte le soin de déterminer la composition qu'elle souhaite pour cette conférence adapté au territoire. Tout en précisant tout de même un certain nombre. De de d'impératif ça dire la représentation des territoires urbains ruraux de montagne ou littorales quand ils existent. Et de lister, à l'image de ce qui existe pour les CIAS ne chers collègues ou les, ou les les CCAS c'est-à-dire c'est la la mairie ou l'intercommunalité qui fixe la composition par contre elle un certain nombre de représentations d'associations ou de structures qui sont obligatoirement. C'est la même logique et ensuite libre à à à à la région de fixer sa propre représentation. C'est un amendement qui ressemble un peu à ce, à ceux qui seront présentés tout à l'heure par Madame Gatel et Madame Cukierman, mais je ne veux pas déflorer le le leur projet qui me semble-t-il, un peu plus simple puisqu'il évite. De, d'avoir à repasser par le vote de l'ensemble des des collectivités. Donc c'est un amendement de souplesse et d'adaptabilité de différenciation. Vial, Monsieur Dantec. L'amendement suivant le 190. Oui, merci Monsieur le Président. Au-delà de la de la forme de cette commission, il y a la question du titre et sur le dit je pense qu'on on fait. À mon avis une erreur en le limitant. Ozanne et à l'artificialisation. D'abord ça risque d'être une commission un peu plus défensive. C'est un peu le sens des débats de. Qu'on a eu. De, depuis le début et alors que. C'est cette conférence Scott même largement ouvert au-delà des Scott hein je reprends pas le le débat, elle va avoir d'autres sujets. Comme dirait Jean Baptiste blanc, c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire c'est que demain, il faut une trame verte et bleue des corridors de biodiversité qui soient efficients, à l'échelle de la région. Demain, cette conférence elle sera obligée d'avoir une vision partagée de l'aménagement du territoire. Et tout cela se retrouve dans le Scott, qui n'est pas que le document lié aux Anne qui est un document qui décline beaucoup d'autres. Politiques publiques donc je pense que rester sur un titre totalement lié. Aux années à l'artificialisation la réduit et peut donner une fausse image de ce que sera son rôle demain alors que c'est une commission, quelle que soit sa composition qui aura un rôle stratégique en termes d'aménagement du territoire et surtout les grandes questions régionales. Merci. Ensuite, deux amendements identiques, le 1er des 2 Madame Gatel le 10 rectifié. Si Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, madame la présidente. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, je l'ai un peu dévoilé tout à l'heure, c'est-à-dire je pense qu'au Sénat. Nous sommes extrêmement respectueux de la libre administration des collectivités de la capacité des collectivités à s'organiser pour prendre en compte la diversité de leur territoire, donc il ne s'agit pas de donner le pouvoir à la région mais de permettre qu'il y ait une proposition d'accord local formulées par le conseil régional mais qui soit naturellement élaboré en accord avec les communes qui ont gardé leur compétence urbanisme ou les interco qui ont la compétence PA lui et que cet accord local soit soumis à l'approbation de ces communes et de ses Interco dans un délai raisonnable qui ne retarde en rien le process de mise en oeuvre Dusan et si dans ces délais impartis, l'accord local n'est pas possible. Le principe défini par la loi et présenté par la présidente et le rapporteur s'appliqueront. Je vous remercie.

De la capacité à pouvoir trouver des accords locaux sur les territoires et une finit d'apporter des réponses si tenté qu'il ne pouvait pas y en avoir De la même façon que nous avons un document identique. Vous me permettrez de citer Madame Gatel en disant que toutefois néanmoins est-ce. Pendant, il a excellemment défendu par elles-mêmes et que donc pour le nôtre il est défendu. Ensuite le 203 rectifier monsieur Corbizet.

En effet celui-ci intègre l'ensemble des normes supérieures que les PLU doivent respecter. La loi notamment inciter les élus à recourir à ce document de planification en fixant une règle d'urbanisation limitée qui s'applique en son absence. Ainsi 97% de la population a 86% des communes françaises sont couvertes par un Scott. Ce qui a permis de réaliser une baisse de 30% de la consommation foncière passant de 30.000 à 20.000 hectares en moyenne par an entre 2011 et 2021. Alors que dans le même temps les communes relevant du règlement national urbanisme ont consommé près de 30.000 hectares. Le présent amendement vise à respecter la place la représentativité des élus travaillant sur la stratégie territoriale des spots, à savoir les EPCI les communes dotées d'un document d'urbanisme mais non couverts par un Scott et cela au sein de la confusion. Conférence régionale gouvernance il invite ainsi la sur-. Représentation d'un même territoire et en particulier des territoires qui ne sont pas dotés d'un du coup du commando urbanisme qui aura pour le ne sont pas concernés directement par la loi. Merci. Ensuite les trois amendements qui suivent sont identiques. Le 5 rectifier bis Madame Gatel. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Il me semble, compte tenu de la taille XXL de certaines régions que les départements ont un rôle d'appui et de conseil à apporter et que donc la proposition suivante qui est celle du groupe de l'Union centriste, consiste à supprimer le rôle uniquement consultatif. Des départements. pour faire en sorte que les départements. Soient associés aux travaux de la conférence, pas à titre consultatif, mais pour un réel avis au regard des compétences que sont les leurs en matière de. De solidarité territoriale d'équité territoriale et en matière également de de préservation des espaces naturels sensibles ou Ile-Rousse joue un rôle majeur. Merci. Ensuite le 167 rectifié. Allez-y, chers collègues. Oui c'est un amendement de Madame Darcos. Ma collègue donc les départements sont des acteurs impliqués dans l'atteinte des Objectifs du zéro artificialisation nette. Il y a plusieurs exemples. L'exemple de l'Essonne par exemple qui a adopté à la fin de l'année 2020 des orientations en matière de lutte contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, pour contribuer à l'objectif zéro artificialisation nette d'ici 2050 en lien avec les partenaires locaux. Cette politique comporte une centaine. Une cinquantaine d'actions pour un budget annuel de un million neuf d'autres exemples que je ne vous proposerai pas. Mais ces exemples de politique conduite sur le terrain prouve que ces collectivités territoriales peuvent jouer un rôle actif au sein de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols. C'est la raison pour laquelle il est proposé qu'il en soit membre à part entière et qu'ils ne soient pas réduits à un rôle consultatif. Telle est l'objet de l'abonnement. Je vous remercie. Allez-y monsieur Brisson. Ce sera. Merci Monsieur le Président. À ce stade où le débat il faut je crois. Trouver un système souple de concertation et d'associations, des élus qui allie proximité vision régionale dès le sens en tout cas ne sait pas sur cet article 3 qui crée la conférence régionale Dusan dans ces conditions, il me semble essentiel de rendre possible quand cela sera nécessaire. L'organisation de cette conférence, sous une forme ou départementales. fait l'étendue du périmètre régional rend difficile l'accès aisé des maires et des élus locaux à cet outil de médiation où il leur sera difficile de défendre les problématiques qu'ils rencontrent dans leur commune garantir aux élus locaux d'accès simple et faciliter à cet outil de médiation et dont l'objectif de cet amendement qui vous propose de permettre une réunion à l'échelon départemental pour tout sujet de réduction d'artificiel sont des sols d'ampleur communal ou intercommunal l'organisation départementale permettra aussi de faire remonter à la conférence de gouvernance, régionale, des analyses et des propositions utiles sur la mise en oeuvre local des objectifs de réduction de l'activité essaieront des sols télé le sens de cet amendement. Merci monsieur Étienne Blanc, le 8 rectifié. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre. Madame, monsieur. Les rapporteurs. En 2 mots. Et le risque c'est que la conférence régionale de gouvernance. Peut conduire à une forme de renversement dans la hiérarchie des normes. le Strada tu dois rester comme le prévoit la loi climat et résilience le schéma stratégique. Et qui permet de territorialiser des trajectoires et d'arbitrer les divergences et les concurrences territoriales éventuelle. ce qui est le proposer cette par cet amendement. C'est de rappeler que la conférence régionale de gouvernance de la politique. Et de réduction et d'artificialisation des sols sera chargé de veiller. À l'intégration et à la mise en oeuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation nette des sols pour éviter cette inversion de la hiérarchie. Et ensuite le 53 rectifié. Qu'il présente Madame Ract-Madoux n'est pas là si si le pardon, excusez-moi. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'avoue que cet amendement et dans la suite mais en fait il a pas beaucoup de rapport hein par la conférence régionale de gouvernance. Cette PPL alezane. Que nous étudions constituent de réelles avancées et je remercie la présidente et le rapporteur pour le travail effectué. Nous savons qu'il faudra gérer 3 périodes pour l'application Dusan. Une avant 2031 une entre 2031 et 2050 et une après 2050 et que ces périodes ont leur spécificité. Nous savons également que tout n'est pas résolu. Cet amendement vise à créer un bilan d'étape dans 5 ans, qui permettra d'évaluer la mise en oeuvre Dusan et ses premiers effets. Et dans ce cadre il paraît nécessaire de prévoir une évaluation à l'horizon 2027 pour 2 raisons et je m'en explique. D'abord la première période déjà entamé des 10 en 2021 2031. Les documents d'urbanisme contraint pas heure de délai d'élaboration seront révisées plus ou moins tardivement par rapport à l'échéance 2031. Ainsi, le risque sera élevé que le foncier. En amont. Donc depuis 2021 de l'approbation des documents dépasse les objectifs de la loi climat résidence l'objectif de 50%. Et impose d'adopter des documents qui devront interdire toute urbanisation mettre un point d'étape. Peu ou prou avant cette date permettra de mieux anticiper les éventuelles difficultés ensuite à partir de 2031 la consommation d'espace entrera dans un système à l'envers le un pour un plus figé et. Qu'il le deviendra à mesure que les friches et de renouvellement densification auront été réutilisés. Il est indispensable que d'ici là les. Les des évolutions puissent être identifiés et qu'on puisse mettre en place. Ces évolutions, il est absolument pas question de remettre en cause Lausanne ni le principe de réduction. On demande juste. La mise en oeuvre de ces aspects quantitatifs Dusan pour. Et et présenter le bilan d'étape. Qui sera remonté par les conférences régionales de gouvernance. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Sur c'est 11 amendements.

Même si c'est un amendement qui inspire un peu ce qui suivent, donc c'est pas un total désaveu. Cédric Vial. C'est même très inspirant. Comme amendement bref. Les amendements Donc que je viens de de citer identique. Prévoit donc que par accord entre la région et les EPCI les communes concernées. C'est par là que soit définie cette composition. un amendement qui poursuit donc l'objectif de précédents que je viens d'évoquer aussi de monsieur Vial, je suis d'accord avec l'objectif donc mesdames. Gatel Cukierman qui relève d'un principe de subsidiarité auquel nous sommes tous très attachés ici ces amendements ont pour nous pour la commission je pense un intérêt qui celui de déterminer la composition par consensus. L'amendement 203 monsieur Corbizet propose de recentrer la conférence sur les représentants des Scott en excluant les représentants des communes ou EPCI, qui sont compris à l'intérêt d'un Scott. Mais l'objet de l'article 3 est bien de permettre aux élus de mieux se faire entendre, car eux aussi devront modifier leurs documents d'urbanisme et à mettre en oeuvre. Je demanderai donc le le retrait des amendements 76 et deux 203 au profit des des amendements 10 et sans. En ce qui concerne l'amendement 190 de monsieur qui propose de maintenir l'appellation conférence et Scott difficile à comprendre qu'l'article 3 instituts bien une concertation avec l'ensemble des parties prenantes bien au-delà des Scott ça sera défavorable pour ces ces raisons-là et je maintiens mon sens de l'histoire pour autant que je partage avec vous Sharon Ronan. En 3ème lieu, certains amendements proposent plutôt des ajouts dans la composition de la conférence régionale. Je veux d'abord rappeler à titre principe que la conférence régionale réunit les autorités compétentes en urbanisme sur toutes les questions relatives à la mise en oeuvre des objectifs de réduction afin d'en débattre et la région il y a donc pas lieu dans les temps de la composition à différentes catégories d'organismes que les collectivités connaissent et consulte. Par ailleurs, même si là aussi c'est le sens de l'histoire, à un moment donné on aura on élargira de toute évidence. En ce qui concerne les associations ou la société civile mais nous sommes là d'abord pour régler les problèmes des élus locaux. Au moment où nous nous nous parlons. il y a trois amendements identiques de nouveau Madame Gatel madame bonne foi Madame Darcos ce qu'il propose que les départements participent à la conférence avec voix délibérative et ce sera un avis favorable à ce titre l'abondement de Monsieur sec Également favorable parce que c'est une idée qui me paraît intéressante, c'est l'amendement 53, Madame Ract-Madoux. Favorable également car il me paraît intéressant et permet de créer en ce sens, qui permet de créer un rendez-vous parlementaire quelques années avant la fin de la première tranche et décennale. Il pourra s'agir de prévoir une transmission au Parlement du bilan que les conférences régionales auront. Réalisé. Et enfin le numéro 8 8, Étienne Blanc qui revient pour. Nous sur le droit existant, puisqu'il supprime la vie que dans. D'ores et déjà la conférence et Scott sur la territorialisation des objectifs qui supprime également le bilan que doit remettre à la conférence régionale de gouvernance. Pour prévoir la place une mission de veille à la place une mission de veille au total, il semble que la proposition de loi propose aussi une définition précise des missions attribuées à la conférence régionale j'en j'en demanderai donc le retrait.

200 398. Le ministre. Si une partie de ces amendements sont adoptés à la fin on pourrait se demander si ça ne veut pas le coup de créer une c'était AP qui associerait l'ensemble des exécutifs à une échelle régionale pour devenir l'instance de discussion, notamment si vous réintégrer les départements. Et j'avoue que le principe qui consiste à dire, chaque région. Pour savoir quelle est la composition de sa conférence régionale Dusan mais vous devez inclure les départements alors même qu'il y a un principe de souplesse sur le fait de voter au moment où vous allez additionner ces mesures. Je pense qu'il y a quelques petits sujets de conformité. Que les obligations de transmission, elles vont se heurter à d'autres dispositions. Le Parlement doit recevoir tous les 5 ans. Le bilan de la loi climat et résilience. Les présidents d'EPCI doivent tous les 3 ans indiquer où ils en sont sur les trajectoires d'artificialisation. Et les conférences des Scott. 3 ans après s'être réunis pour la dernière fois tu doit faire le bilan de la où en sont les trajectoires. Nous rajoutons en quelque sorte avec cette conférence des ânes. Un nouvel échelon de transmission qui va s'ajouter à un échelon intercommunal et un échelon national. Sagesse. Bien, donc nous allons avis de sagesse sur l'ensemble des amendements du gouvernement. Je vais les soumettre aux voix dans l'ordre où ils ont été présentés en vous rappelant à chaque fois l'avis de la commission. Donc. Et en en demandant aux auteurs. Si les rôtir là où ils sont, monsieur Vial. Puisque c'est le premier le vôtre justement

la rédaction de mon amendement permettait un peu plus de souplesse et évitait d'aller chercher des délibérations dans l'ensemble des collectivités. Qui ont la compétence urbanistes donc PLU Hooper lui donc ça me semblait un peu plus souple et un peu plus simple. je m'excuse auprès des 37 co-signataire de cet amendement mais je me fie à la sagesse du rapporteur, et je retire cet amendement. Donc le 76 et retirer ensuite le 190 si un avis défavorable de la commission sagesse Monsieur Dantec. Je vous le maintenez. Donc il est soumis, on voit avec un avis défavorable de la commission, la sagesse du gouvernement le 190. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Ensuite, on a 2 amendements identiques, le 10 et le 111 avec un avis favorable de la commission David. Pardon.

Les contre. Qui s'abstient. Ils sont adoptés, ensuite le 203, une demande de retrait de la commission. Donc qu'il est maintenu. Non il est retiré. Il est retiré. Ensuite on a trois amendements identiques, le cinq, le 125 et le 167 avec un avis favorable de la commission. Et est toujours avide sagesse du gouvernement qui est favorable. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils sont adoptés. Ensuite, un avis favorable sur le 59 de la commission avis de sagesse du Gouvernement toujours qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Une demande de retrait pour le huit Monsieur Étienne Blanc il est retiré et un avis favorable sur le 53. Qui est de la commission a vite sagesse du gouvernement qui est pour le 53. Qui est contre. Qui s'abstient il être adopté. Voilà donc pour c'est 11 amendements, nous passons. Ensuite à 2 amendements en discussion commune le 214 Madame Gacquerre. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement vise à introduire une représentation des professionnels du logement et notamment du logement social au sein des conférences régionales de gouvernance au regard des enjeux considérables de la mise en oeuvre Dusan en particulier sur les politiques de l'habitat. Le mouvement HLM est un acteur incontournable pour accompagner la petite nation Suzanne dans les territoires pour exprimer les besoins en logements à loyer modéré pour garantir la mixité sociale et l'équilibre entre les territoires au travers de cet amendement. Je souhaite alerter sur les dangers Dusan sur le logement, plus précisément sur le logement social accessible aux Français les plus modestes. Le nombre de ménages a augmenté de 20% en 20 ans. Augmentation qui se traduit nécessairement par une hausse significative de la demande de logement et plus encore de logements sociaux. Parallèlement, l'offre ne suit pas, notamment en raison de la rareté des terrains constructibles en ville et l'explosion des coûts de construction, la mise en oeuvre de l'objectif than risque d'aggraver considérablement la situation, notamment parce que Lausanne va se traduire par une réduction significative du foncier constructible ce qui impactera forcément les coûts de construction et par conséquent pèsera sur la construction de logements. Une question se pose donc aujourd'hui notamment la façon dont le gouvernement va concilier Lausanne avec la construction de logements et notamment de logements sociaux hein des. Indéniablement, il va falloir penser un nouveau modèle économique qui nous amènera repenser la construction la densification et l'aménagement de l'espace. Autre sujet logement important la mise en oeuvre Dusan qui menace la pleine application de la loi SRU qui impose aux communes de plus de 3500 habitants appartenant à un et un EPCI de plus de 50.000 habitants de disposer de 25% de logement social, d'ici 2025. En l'état, cet objectif n'est pas conciliable avec Lausanne et constitue un casse-tête pour les maires et pour les élus locaux sur ce point également un éclaircissement du gouvernement sur l'adaptation de la loi SRU aux objectifs Dusan nous semble nécessaire pour finir et pour toutes ces raisons, l'intégration des acteurs du logement, notamment du logement social s'avère indispensable dans la mise en oeuvre Dusan afin de garantir une réponse adaptée aux besoins logement que connaît notre pays. Il s'agit ici de l'objet de l'amendement que je vous propose, je vous remercie. Merci et ensuite en discussion commune le 248 Monsieur Bonhomme. Merci monsieur le président. Toujours dans le cadre de cette mise en oeuvre. De la politique de réduction de l'artifice ceux des sols. Les conférences régionales de gouvernance doivent au pouvoir à titre consultatif, s'appuyer sur l'expertise des professionnels de l'aménagement et de la construction qu'on soit architecte urbaniste ou encore paysagiste, concepteur en effet les intégrer au dispositif permettrait aux élus, représentants des collectivités locales de bénéficier de plusieurs plus-values notamment leur analyse sur les projets en cours et sur les difficultés rencontrées sur le terrain pour atteindre l'objectif de sobriété foncière ou encore d'avoir un éclairage sur les questions liées au marché immobilier à l'évolution de la demande des ménages. Et également. De bénéficier de d'éléments opérationnels sur par exemple les potentialités de la compensation selon les spécificités de chaque territoire et d'avoir une photographie plus précise des acteurs locaux sur lesquels ils peuvent s'appuyer De se voir proposer une analyse de l'impact du sur l'évolution des prix du foncier. Vous savez qu'en ce moment et pour les années à venir la la question du logement, de la crise du logement qu'on nous annonce et qui arrive de contenu de détention qui a sur le marché de l'offre et de la demande de logement. Ce serait un élément important me semble-t-il cette possibilité cette intégration donc, des représentants des professions de l'aménagement. Sur le terrain paraît pertinente. Au regard de l'objectif de donner un caractère opérationnel l'objectif Anne. Merci Monsieur Bonhomme avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Sur ces deux amendements. Monsieur le président. Sur ces deux amendements. Ça aurait une demande de retrait sinon défavorable. Alors ce sera la même position concernant les amendements qui qui est, savoir que bien bien sûr se ces arguments sont intéressants et et légitime, mais nous avons voulu une conférence régionale sur une conférence d'élus d'autorités locales compétentes en matière de d'urbanisme. Pour ces raisons là ce sera donc bien un retrait sinon défavorable. Monsieur le ministre. Merci monsieur le président. Plusieurs éléments. D'abord sur les logements sociaux. L'artificialisation a progressé de 70 pour 140 ans, la population de 20%, qu'il aurait un lien automatique entre le foncier disponible et la disponibilité pour le logement en particulier sociale ne tient pas. D'autant plus que 84% des logements sociaux dans ce pays sont des collectifs. La part de logement social en maison individuelle est plus faible et donc la diminution potentielle du foncier disponible. N'aurait pas d'impact, on soit sur le logement social, le sujet c'est la volonté des élus et la disponibilité, commune par commune du foncier disponible. De ce point de vue, vous avez déjà avec la loi 3DS modifier une partie de ce que sont les objectifs de la loi SRU et ce que je pense fondamentalement c'est que s'abriter derrière Lausanne pour expliquer qu'on ne peut pas tenir une trajectoire de construction de logement social, c'est un prétexte. Sinon toutes les communes à la minute où on se parle aurait déjà suffisamment de logements sociaux, on a des communes qui ont foncier et qui ne font pas et on a des communes qui veulent faire mais qui n'ont pas le foncier, mais dire que c'est à cause du Dusan ça n'est pas exact, et tous dans nos départements, nous connaissons. Des communes qui sont dans des situations qui sont diverses, où tout ne s'explique pas par la disponibilité ou l'indisponibilité de foncier, je le redis. Le logement, ça peut être le cas parfois, mais à ce moment-là, on est davantage dans la loi 3DS. Ils ont les assouplissements qui viennent d'être votées, qui commence à s'appliquer pour partie cette année et donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les 2 sujets en particulier parce qu'on a cette problématique est une problématique collective. Ensuite. Plus largement sur l'association des uns et des autres. Je vais rester sur une position de sagesse, mais ce qui m'embête si vous le votez si vous votez ces deux amendements. C'est que pourquoi ce qui serait vrai. Sur l'artificialisation ne le serait pas sur les Scott sur les plus et sur un certain nombre d'autres documents d'urbanisme ou l'avis des professionnels et du mouvement social pourrait à ce moment-là se justifier pour les mêmes raisons. Puisqu'à la fin la typologie de ce qui se construit, où la nature des concertations qui sont conduites elle mérite ce regard d'expert. Ce serait faire injure aux élus locaux, que de penser que eux-mêmes ne s'entoure pas de ce type de conseil pour élaborer leur Scott ou leur plus. Ou même pour avancer sur des opérations. Donc je reste sur une position officielle de sagesse mais je pense que si on met le doigt là dedans. Ensuite ça conduira à modifier les échelons communaux et intercommunaux de prise de décision sur le plan de l'urbanisme et que ça nous entraîne sans doute à un endroit où on n'a pas collectivement envie d'aller. Donc on a plusieurs demandes de prise de parole Madame Lienemann. Je partage avis de la commission sur le fait que c'est difficile d'introduire les professionnels du logement dans ce genre de structures en plus lesquelles les bailleurs est bailleur. Quelle. Qu'elle. L'UNPI, bon bref qui ont mais déjà c'est un 1er problème. Néanmoins il est clair que Lausanne va poser de lourdes difficultés. Pour atteinte des objectifs de construction de logements et de rénovation restructuration de logements dans le pays a besoin. Et il y a un impensé total qui a l'effet prix sur le foncier. Et à partir du moment où on a une rareté. Il a pas besoin des, des grands spécialistes du marché pour savoir que tendanciellement, ça va augmenter les prix du foncier. Or on a déjà pour boucler les opérations de logement social. Voix et qu'elle soit d'ailleurs en locatif ou en accession sociale à la propriété mais même parfois pour du logement intermédiaire d'immenses difficultés aujourd'hui à. Boucler les opérations. Donc s'il n'y a pas une politique de régulation des prix du foncé. Pour éviter une hausse et pour mieux encadrer les évolutions. Vous allez avoir inéluctablement premièrement une réduction de la production, mais surtout une éviction de du logement, le plus abordable pour nos concitoyens et ça c'est, de mon point de vue là, une des questions majeures qui se pose devant nous. La 2ème c'est que même si le vous réduisez le foncier, la mutation faire muter la ville sur la ville où le bâti sur le bâti coûte bien plus cher que quand vous faites sur du neuf et on a le même problème. Cette décision rendra plus coûteuses les réalisations de logement. Je ne crois pas que la nation est pris la mesure de ce que ça suppose soit d'implication publique soit de régulation des prix qui en matière de foncier est tabou depuis des années, des années et amène à fait que dans notre pays le foncier a augmenté plus que tout autre chose. Plus que les salaires plus que les placements. Productifs. Bref, c'est aussi une rente injuste. Merci cher collègue. Madame Gatel. Sous le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente. Monsieur le rapporteur. Moi je suis j'en j'entends et je suivrai. L'avis du rapporteur sur l'amendement notre collègue hackers mais toutefois je tiens la tension comme notre collègue l'a fait sur le fait et le ministre a raison, ça n'est pas Lausanne qui va empêcher la construction de logements sociaux mais il ne va pas forcément aidé à cause de la spéculation et je voudrais citer l'exemple d'une commune de Loire Atlantique et Le Croisic. Touché par la loi littoral. Il aurait su 1000 m2 de terrain impossibles qui appartiennent un particulier. Alors même qu'elle a l'obligation de construire des logements sociaux. Donc Monsieur le Ministre, vous avez raison, moi je pense qu'il faut activer ce que nous avons défendu avec notre collègue avec nos collègues d'Arnaud Estrosi Sassone et Valérie Létard sur 3DS, avec ce contrat de mixité sociale, qui encore une fois, permet de faire valoir le pouvoir réglementaire locale intelligent d'un préfet intelligent. Qui prend en compte la situation, la bonne volonté des maires et parfois l'incapacité. Donc je vous rejoins et je pense que c'est. Une bonne idée, Monsieur le Ministre, de vous rappeler de 3 DS c'est pas mal ça. ça. Calcaire. Merci, monsieur le Ministre, j'aimerais revenir sur ce que vous avez évoqué, la première chose concernant ce que vous avez évoqués sur le Lausanne qui serait un prétexte pour les mères de ne pas construire de logements sociaux. Je vous trouve très dur. Vous avez été maire. Je pense que les maires assument leur décision n'ont pas besoin Dusan pour avoir ce prétexte là, aujourd'hui, les maires ont envie de construire parce qu'ils ont envie d'héberger de trouver des logements de proposer des logements à leurs habitants et à tous les habitants, notamment ceux qui aujourd'hui des revenus modestes. Ça c'est la première chose et la 2ème. Ce que je disais c'est cuit Lausanne va complexifier la construction de logements sociaux, c'est une réalité. Le prix du foncier a déjà commencé à augmenter. Il va exploser. il a explosé et il va Poutine donc non. Oui pardon ça va complexifier en tout cas la construction de logements et puis j'aimerais terminer par une chose qui est une réalité, c'est que là aujourd'hui on a quand même 1,7 millions de demandes de logements sociaux qu'qui n'est pas à laquelle on ne répond pas donc il y a une vraie demande et donc il y a nécessité de construire et comme le le le le modèle économique n'est pas qu'on soit aujourd'hui on va devoir réinventer hein ça va devenir très complexe. Donc c'est un vrai sujet sur lequel on attend une réponse de votre part, je vous remercie. Madame la présidente. Et ensuite, Monsieur le Ministre, madame la présidente. avec ma collègue Dominique Estrosi. Avec ma collègue Marie-Noëlle Lienemann hé bien des élus ici est au coeur de nos préoccupations au coeur de nos préoccupations et Viviane qui est là-bas. Simplement. On parle d'un amendement qui revient à proposer de mettre l'FPI et le FSB dans la gouvernance décentralisée Dusan et donc on peut partager ça et les difficultés qu'a évoqué Amel Gacquerre. des conjonctions en fait. D'obligation d'injonction donnée aux territoires d'être au rendez-vous de la production de logement social et on ne peut pas s'y opposer mais dans le même temps de dire on va vous mettre une pression foncière supplémentaire qui va renchérir les coûts. Encourager à la requalification des friches qui va augmenter encore l'impact sur la production de logement social, tout ça est compliqué, mais le sujet et j'attire votre attention que nous devons voter c'est est-ce qu'on met la FPI et la FSB dans la gouvernance territoriale. Je pense que non, je pense qu'il faut être prudent, c'est la gouvernance décentralisée Dusan elle concerne les collectivités. C'est comme si on mettait un promoteur immobilier dans les conseils municipaux. Voilà, pour être clair. Monsieur le Ministre. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour répondre à la sénatrice gars car je vais faire par anticipation la pub de mesures proposées par Valérie Létard et Jean-Baptiste Leblanc. Parce que dans les outils que vous allez proposer sur le droit de préemption sur le sursis à statuer. On a des mécanismes qui vont permettre d'éviter une spéculation un phénomène de rente. Ça c'est le 1er niveau il y a 4 ou 5 dispositifs et je les soutiens. Pour cette raison et le gouvernement les encourage parce qu'ils pensent qu'ils peuvent permettent de corriger ça. Ensuite. Mais c'est pas l'objet de la discussion de ce soir il y aura le volet financement. Moi je suis sensible à ce qu'a dit Madame Lienemann et à la fin on ne peut pas avoir un phénomène dans lequel on va chercher de l'argent public pour dépolluer les friches sans se préoccuper de la manière dont on renchérit en quelque sorte pour le promoteur, le coût de l'artificialisation si on juge que c'est pas souhaitable et on peut avoir une conjonction entre les deux, c'est qu'une part de la rente qui soient générés par la rareté qu'on a. Produite. Elle alimente. Les recettes des collectivités territoriales pour leur permettent d'aller chercher les recettes qui leur permettent d'accompagner le dispositif parce que si je dis à moins de foncier disponible. Je crée un effet de valeur supplémentaire par rapport à la valeur normale. Et donc je suis une rente qu'une part de cette rente revienne à la collectivité. Ça ne me choque pas, ça n'empêche pas celui qui vend son terrain agricole de faire un foie 30 mais cela permet à la collectivité de récupérer des crédits qui lui permettent de conduire une politique sociale. que ce sera l'occasion sans doute de parler de bail réel solidaire d'office foncier de PF de beaucoup de dispositifs qu'on a mis en place qui ne sont pas forcément utilisés et qui m'ont conduit à dire que dans le lot, ma formule était peut-être brutale mais. Il y a de tout, on a des élus qui sont dans une vraie incapacité. On en a d'autres qui utiliseront ce prétexte, en plus de doutes qui utilise parfois déjà. Ensuite, c'est la démocratie qui s'applique, c'est la réalité des 1000 communes dans notre pays qui ne respectent pas le rue il y en a qui cherche les moyens il y en a d'autres qui ne les cherchent pas. Ces. Monsieur Richard. Ce sera court, Monsieur le Président, je ne voterai pas ces amendements pour les raisons qui ont été indiquées. Mais je dois dire très franchement que les explications de Monsieur le Ministre ne m'ont pas convaincu. Moi je suis effectivement persuadé comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure que Lausanne va rendre plus difficile plus difficile la la la la possibilité pour les communes simplement de s'acquitter à leurs obligations en matière de logement social lorsqu'elles ont plus de 3500 habitants inclus dans une. Intercommunalité de plus de 50.000 ça va rendre plus difficile plus compliqué. Monsieur le Ministre, quand vous leur dites charge pour elle d'aller chercher l'argent c'est déjà c'est déjà un aveu de la difficulté de la complication que vous leur vous vous le remettez en en charge. On le voit bien, si c'était facile, au jour d'aujourd'hui je je mets de côté

on les sanctionne financièrement et caetera, le contrat de mixité sociale le 3DS doit faciliter les choses, c'est sûr, mais malgré cela, ça va encore une fois ça va renchérir les coûts à non pas douter ça va renchérir le coût. Vous venez de le dire, vous-même pour trouver effectivement des solutions financières leur permettant de de de réaliser quand même je le répète vous compliqué avec Lausanne. La situation de ces communes et personnellement ce n'est pas acceptable. ou alors encore une fois. Proposez heure un outil leur permettant effectivement de de de de de de passer. Outre ces complications telle façon à ce qu'effectivement l'objectif attendu par tout le monde puisse être atteint.

Qui est contre. Qui s'abstient ou pas. Adopté ensuite l'amendement 248 de Monsieur bonhomme avec un double avis défavorable également il est mort. Ensuite, nous passons à l'amendement 221 monsieur Corbizet. Oui, merci Monsieur le Président. C'est vrai que le développement urbain. Durable ne doit pas entrer en concurrence avec les besoins de. De logements. En particulier des plus modestes Mac l'Anita Kerr si elle m'écoute effectivement a raison c'est 1,7 millions de personnes qui sont en attente d'un attribut d'attribution d'un logement social. Or mutation.

alors que nous sommes en retard sur la production de logements sociaux. Lausanne va freiner effectivement cette capacité de production de chance de qualité. C'est pour ça que moi aussi je souhaitais que les organismes du mouvement HLM et uniquement HLM pour pas qu'effectivement il y a des spéculateurs soient présents au sein des conférences régionales gouvernance

Or, quand on a besoin de populations. En centre-ville on on préfère construire de du logement en se retrouver le prêtre proche des des commerces et des services municipaux. J'entends Madame Lienemann qui me dit oui mais restructuré centre-ville ça va coûter plus cher que de construire à l'extérieur donc en gros on va. Inciter les communes à consommer des Terres agricoles pour faire du logement en dehors de la ville et non pas sur le curé le le le le bâti ancien dégradé pour refaire de du Alors ah ça sert à quoi l'ANRU là où il y a quand même été là pour un moment donné et des des collectivités pour restructurer de de l'habitat ancien, et de ne pas consommer des Terres agricoles. Donc j'avoue un moment là ne le les perdre un petit peu. Monsieur le Ministre, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné on va être en très grande difficulté en la matière parce que d'un côté on nous venez à vous dire avec le climat. La loi climat madame Pompili. Il faut mettre de la verdure dans les dents creuses alors qu'on pourra faire. Bâtir. Je rappelle que dans les Scott, on vous incite à construire plus une dizaine de logements par an

une zone de vie ailleurs donc parfois construire sur des Terres agricoles, ça peut coûter plus cher que dans le le centre-ville et le mouvement HLM, c'est faire en centre-ville. Je vous remercie. Monsieur le président, ce sera pour les mêmes raisons que je demanderai. Un retrait sinon défavorable. La France. Monsieur le ministre. Même avis monsieur Corbizet si vous le maintenez. Oui. Donc, je le soumets aux voit avec un double avis défavorable 221 rectifié qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté ensuite trois amendements identiques. Le 34 rectifié, monsieur, bonjour. Monsieur le président, monsieur Miss monsieur madame la présidente. Monsieur le rapporteur. La conférence régionale de gouvernance auront notamment pour mission de rendre avis sur l'inscription dans les sera des projets prévus par les articles 4 et 5 de la présente, proposition de loi. Parmi ses nombreux projets, ce qui présente un intérêt majeur pour les acteurs économiques des territoires voir sont portés directement par ces acteurs. C'est le cas notamment des implantations d'unités industrielles valorisant l'utilisation d'une ressource naturelle renouvelable concourant à la transition énergétique ou relevant de l'indépendance nationale critères prévus par l'article IV. Dès lors, il est important que ces acteurs économiques puissent s'exprimer lors des discussions prévues par les conférences régionales de gouvernance cet amendement propose donc que ces conférences ouvertes à 6 représentants des chambres consulaires. Qui vous remercie. Oui, monsieur le président. Merci Monsieur le Ministre, mes chers collègues ont c'est un amendement identique effectivement les acteurs économiques sont complètement partie prenante de l'aménagement de nos territoires. Il paraît normal qu'il puisse être associés aux conférences de gouvernance. Merci. Merci et le 105 rectifier bis monsieur Jeannet merci, monsieur le président. Mais. Collègues viennent de défendre excellemment cet amendement peut être rajouter quand même à nouveau le constat concernant. Le lien entre cette politique de ans et les politiques de développement économique en particulier. Peut être appelé également le constat. Toutes activités confondues, la part du foncier économique dans les surfaces urbanisées est en baisse depuis ces 10 dernières années, mais depuis 2 ou 3 ans, nous observons une hausse de la demande foncière pour les autres activités industrielles et logistiques sous l'effet du E-commerce et de la réindustrialisation, dont on peut espérer qu'elle s'amplifie ses activités nécessitent des espaces de stockage important pour entreposer des biens des matériaux, ce qui demande en général beaucoup de de foncier. dit à propos du logement mais effectivement cette concurrence entre les implantations d'activités et la production de logements à l'heure Dusan ne peut que. Et donc. Effectivement ça fait apparaître un certain nombre de crainte aujourd'hui sur un bon nombre de territoires concernant ses implantations d'activités économiques. Rajouter à cela que par exemple les évolutions fiscales avec la suppression des impôts de production. Avec des évolutions sociétales et également qui font que parfois, certaines activités industrielles sont désormais difficile à implanter sur notre territoire, parce que vous avez toujours des opposants qui préfèrent le. Effectivement ne pas avoir. De d'activité. À leur porte et donc je crois qu'il faut avoir en tête que l'ensemble de ces politiques ne doivent pas dissuadé aux implantations ne doivent pas dissuader les élus de renforcer les capacités d'accueil de ces activités économiques. C'est pourquoi la présence des. Des chambres consulaires régionales au sein de la confessera. Conférence régionale de gouvernance apparaît tout à fait opportune. Merci monsieur le rapporteur. Sur ces trois amendements identiques. monsieur le président. Chers collègues, sur ces trois amendements, alors c'est toujours la même question hein. On propose une conférence régionale de Dusan cette conférence décentralisé. Donc c'est une question d'élus encore une fois, nous cherchons des outils pour les élus locaux pour appréhender la trajectoire Dusan faut-il ouvrir non seulement à des associations ma des représentants du monde HLM ou à des CCI. C'est une question en effet. Je n'ai absolument rien contre les CCI. Par ailleurs, je précise. Et donc mais c'est une première question que nous devons trancher, est-ce que des CCI sont en charge de l'urbanisme, il me semble que non développement éco bien sûr mais voilà, ce n'est pas strictement de de l'urbanisme et puis un tout petit détail qui n'en est pas hein. Chers collègue participation de 6 représentants des CCI, c'est-à-dire plus que les élus. Donc ce sera une demande de retrait sinon défavorable. Monsieur le Ministre. Défavorable sous l'angle effectivement de la confiance aux élus qui sont censés représenter les différents éléments et quelques je comprends les chambres consulaires, ça voudrait dire qu'il y aurait les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie avec à l'intérieur de ces chambres consulaires d'autres débats et je pense que il y aurait une vraie sagesse pour le coup, à rester à l'Inter d'une représentation des élus territoriaux. Il y a un merci président Longeau. Je le retire au vu des s'explications du ministre et du rapporteur. Il a il est retiré. Madame Beyreuther. Monsieur Jeannet. Oui je, j'entends avec beaucoup d'attention les les arguments du rapporteur. Et du ministre. J'étais un peu plus optimiste lorsque le rapporteur avait dit qu'il trouvait tous nos amendements intéressant et légitime. Peut-être quand même qu'il faudrait réfléchir à notre proposition, dans la mesure où justement le fait de mettre autour de la table et Monsieur le Ministre, vous répétiez combien vous étiez intéressé de pouvoir avoir une réflexion au niveau régional pour le pilotage de tout cela qu'au niveau régional, on puisse entendre autour de la table, la voix des différents acteurs économiques et en particulier. Les CCI mais aussi les chambres d'agriculture comme ça vient d'être dit. On on a rappelé que. Une bonne partie de la motivation de Suzanne c'est également de la protection des Terres agricoles, je pense que le dialogue qui pourrait en ressortir serait tout à fait intéressant et peut-être que dans la suite de la discussion parlementaire. On pourrait garder cette idée dans un coin de vos esprits mesdames et messieurs et aussi qu'on pourrait inviter ses acteurs à participer à cette conférence avec un avis consultatif. Sans forcément participer au au vote mais ça permettrait de trouver. Un compromis intéressant pour éclairer utilement les débats. Mais donc je fais confiance au rapporteur pour porter cette idée un peu plus loin et donc je retire. Pour l'instant cet amendement. Bien merci donc les les trois amendements sont retirés. Nous continuons avec la discussion de deux amendements en discussion commune le 124 rectifié madame bonne foi. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à élargir la conférence régionale à d'autres membres que ceux prévus au présent article ainsi. Je vous propose d'intégrer à cette conférence. 4 représentants d'organismes compétents en matière de biodiversité tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux etc 3 représentants d'associations de protection de l'environnement. Quand je pense que la société civile doit avoir toute sa place dans cette conférence, un représentant de l'ARS. Car le sujet de la santé environnementale, la qualité de l'eau doivent être au coeur des préoccupations sur l'artificialisation ainsi en complétant la composition des membres de la conférence régionale par des personnes ayant des connaissances objectives et renseigner sur les questions écosystémique. Je pense que nous pouvons apporter une réelle plus-Value aux futures délibérations de cette. Conférence donc les personnes qualifiées serait un atout considérable pour venir éclairer les décisions des collectivités. Merci et le suivant, Madame Préville. est bénéfique pour la mise en oeuvre de Cezanne dans les territoires. Mais il n'y a pas de représentants d'organismes d'associations compétentes en Gestion et protection des espaces naturels. Si de tels représentants peuvent être consultées, mais le seront-ils leur présence dans la gouvernance Dusan serait tout à fait justifiée en la matière. D'Intelligence collective qui est très précieuse, elle doit pouvoir se vivre et notamment au sein de telles instances car en effet Lusa n'a pour vocation principale de préserver les espaces naturels et leur biodiversité. Il est donc essentiel que des personnes compétentes dans ce domaine puissent participer à ces conférences. On ne peut plus raisonner en silos maintenant siéger ensemble avec des représentants compétents sur ces sujets d'environnement et de biodiversité, me paraît être une amorce d'un véritable changement, chacun pourra se nourrir des autres d'autres points de vue c'est vertueux. Il s'agit de donner une autre dimension à cette gouvernance qui doit faire des choix éclairés la personne la la parole de ces personnes pourraient être très intéressantes. Car, Lausanne. Ce n'est pas uniquement des choix comptables. Il ne peut pas s'agir simplement de questions de superficie et ce serait dommage de louper le coche en en fait d'une gestion différente plus fine qui tiendrait compte de la spécificité véritable de nos territoires et notamment des terrains Merci monsieur le rapporteur. Sur ces deux amendements. Hé bien. Monsieur le président, ce sera aussi. Demande de retrait sinon défavorable pour les mêmes raisons, j'indique toutefois. Un autre collègue que rien n'empêche. La conférence des zones de consulter. Pour avis les organismes mentionnés. Monsieur le Ministre. qui représentent aussi la diversité des sensibilités économiques, environnementales et que de représentativité qui s'affronteraient. Celle des associations et celle des élus ça viendrait considérablement compliqué la tâche après de la région sur la base de cet échelon de concertation. Donc un double avis défavorable sur ces deux amendements. Je les soumets au revoir. Madame Préville. Ce serait juste pour dire que moi je n'ai proposé que 2 représentants donc un représentant d'organismes compétents et 1 représenteront d'association par rapport à la dizaine de personnes élus effectivement ce serait juste pour apporter un éclairage complémentaire c'est tout. Merci. Donc je soumets au voile 124 rectifié qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient et ensuite le 144 rectifié qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté ensuite l'amendement 113 rectifié monsieur ai. Il s'agit d'un amendement qui vise à assurer le respect de l'objectif de recyclage des friches. À l'échelle régionale qui correspond à une échelle de territoires pertinents pour un tel objectif est de rang de la conférence régionale de gouvernance compétente pour son n'application après tout ce que nous venons de dire sur la composition de ces conférences régionales sur leur rôle également. Il apparaît utile ou en tous les cas légitime qu'elle puisse se. Positionner en tous les cas étudiés. Cette problématique des friches puisque souvent dans l'évocation Dusan. sources d'espoir qui nous sont donnés pour que l'artificialisation nette ne conduisent pas à bloquer des projets, c'est d'utiliser. Ces friches mais sur un territoire des problèmes de localisation de pollution et de dépollution. De les enjeux de renaturation également, tout cela peut faire effectivement que. Le recyclage de la friche ne soit pas aussi simple qu'il puisse y paraître. Et donc cette conférence. Est régional de gouvernance composée, on l'a bien compris exclusivement d'élus puissent être sensibilisés à ces sujets, on peut espérer également que dans les avis qu'elle rendrait elle pourrait inciter les régions et les acteurs locaux à aller également sur le financement et sur l'incitation à ces recyclage de friches. C'est un sujet qui mérite certainement qu'on puisse y arrêter quelques instants. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le président, notre collègue Fabien sous mais de nouveau à l'Assemblée une idée intéressante. Toutefois, il nous semble que. Le la conférence régionale va d'abord s'occuper de la trajectoire Dusan. Peut-être que ce cet autre sujet des friches viendra par suite notamment la leur recyclage donc il nous ça semble quand l'état dans le cas cette instance consultative il ne convient pas trop d'en élargir son objet. Ce sera donc un retrait Simon défavorable. Merci monsieur le ministre. Défavorable pour deux raisons, la première c'est pour l'objectif annuel en matière d'aménagement. C'est compliqué de se fixer un objectif annuel lors que parfois, il peut y avoir besoin d'un peu plus de temps particulier pour de la dépollution de friches, même si je partage l'intérêt et ensuite. Moins la région à de pouvoir prescriptif, plus ça devient compliqué de lui demander de coordonner un objectif de baisse des friches donc sans malice. Ce que je dis, c'est que l'objectif, il est très juste, mais qu'à partir du moment où vous avez voté la prise en compte. Plutôt que la compatibilité. On ne peut pas en plus demander maintenant à la région d'avoir une trajectoire annuelle de friches sinon on on on la rend responsable de quelque chose sur lequel la plus la même main que ce qui avait au début du texte.

qui serait de considérer que la trajectoire Dusan. Et peut-être faut-il rappeler à cet instant que zone C zéro artificialisation nette, c'est-à-dire à la fois avec de la, des espaces que l'on pourrait. Consommer d'autres qu'on l'on pourrait rendre aux activités agricoles ou à la à la nature. Forcément, forcément que les friches sont des éléments importants au regard même de ce que représente au niveau national ces surfaces dans la trajectoire du jeune ou alors je n'ai rien compris à tout ce que nous disons depuis quelques jours maintenant que nous étudions cette proposition de loi. Je dois avouer également que pour le coup, et peut être pour une fois les arguments de Monsieur le Ministre. Serait sans doute de nature à me convaincre et qui effectivement la rédaction de l'amendement. En particulier avec le l'objectif annuel semble difficile à. À suivre. Et donc c'est pourquoi. À la fois par respect. Pour le travail et la confiance que j'ai au rapporteur et pour l'argument donné par le ministre, je retire cet amendement. Bien merci chers collègue l'amendement est retiré. Donc je vais soumettre aux voix l'article 3. Qui est pour l'article 3. Qui est contre. Qui s'abstient.-il être adopté. Nous passons à la discussion de l'article IV. madame la présidente, excusez-moi. Il est 23h 22. Juste nous avançons donc à elle au rythme de 10 amendements à l'heure 179 amendements, ça veut dire au même rythme, 18h. Nous n'aurons pas assez de la soirée et de jeudi. dans l'après-midi et la soirée pour venir à bout de l'ensemble des amendements. Donc je vous encourage juste. À bien vouloir essayer de. De réduire peut-être aux explications de vote ou vos temps de parole. Non pas pour vous interdire de vous exprimer. On a eu 35, prise de parole. Avant l'article 1er, il me semble que chacun a eu l'occasion largement d'exprimer de son point de vue au-delà de la digue discussion générale merci. merci madame la présidente. Donc nous. Pour l'heure, nous poursuivons en essayant de ne pas fléchir et l'article IV. J'ai une demande de prise de parole de notre collègue, Béatrice Gosselin, allez-y, chers collègues. Monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, je vais en premier lieu remercier nos collègues, madame la présidente et monsieur le rapporteur pour l'excellent travail très sensible sur les modalités de mise en place de Cezanne. L'obtention d'un décompte spécifique pour les projets nationaux dans une enveloppe distincte de la trajectoire envisagée par le pour le bloc local qui se traduit par un premier effort territorialisée de 50% pour les 10 prochaines années avant le zéro artificialisation nette en 2050 m'apparaît être une avancée importante que je tiens à souligner. De même, il est tout à fait pertinent d'appliquer la trajectoire Ouazzane. À des projets d'intérêts nationaux comme aux autres projets de l'enveloppe régionale ou du bloc local ainsi collectivités et État sont logés à la même enseigne. Pour autant, si la solidarité s'exprime entre les territoires. Avec cette enveloppe et conduit à ce que certains projets consommateurs d'espace et pour autant indispensable reste réalisable. Il importe néanmoins d'être vigilant sur le contenu des projets pouvant entrer dans le cadre de l'enveloppe de ces projets nationaux et de l'encadré par exemple par décret. Car l'objectif étant nationale le compte foncier à partie à répartir entre les régions françaises, sera bien celui déduit de cette enveloppe. Et c'est vrai également par ricochet pour l'enveloppe locales. serait pour il. Il se pourrait que certains territoires ou région puissent être pénalisés parce que l'État aura concentré sur une période donnée des priorités dans un endroit ou à un autre de France sur lequel l'enveloppe nationale sera combien consommer. Je vous remercie. Merci cher collègue. Nous allons donc passer. À la discussion des amendements ont commençons par deux amendements de rédaction globale de l'article. Le 1er présentée par le gouvernement le 181. Monsieur le Ministre. Très bien. Sortir les grands projets de. D'envergure nationale des trajectoires régional, c'est l'engagement qu'Élisabeth Borne a pris. Devant l'AMF à la fin du congrès des maires. Le sujet. Qui rejoint la préoccupation du Sénat. Y compris d'ailleurs avant cette. Officialisation par la Première ministre que nous y étions prêts. Ils se heurtent, maintenant la question de qu'est-ce qu'on met dedans. Et je dois dire que la discussion qui nous attend. Malgré les consignes de Valérie Létard promet sans doute une multiplicité de discussion puisqu'entre les bâtiments agricoles. Les projets qui participe à la transition écologique, les projets liés à l'eau les projets liés aux déchets les projets l'économie circulaire les projets en lien avec la protection des populations et des risques tous les bâtiments publics d'intérêt collectif, les routes départementales les projets portés par les épiques les logements rendus nécessaires par les grands projets industriels les projets de la circonscription portuaire du Havre, les projets inscrits dans la circonscription administrative de tous les ports, les opérations de revitalisation. Les quartiers de gare les quartiers autour des stations de transports publics et les exutoires de déchets du grand Express Paris qui synthétise la quasi-totalité des amendements que vous avez déposé en plus de ce qui est déjà dans l'article. Si on prend tout ça. Je pense qu'on est capable d'artificialiser davantage dans les années qui viennent que ce qu'on a fait par le passé. La proposition du gouvernement les triple. Elle consiste à dire dans le texte on assume de sortir les grands projets d'envergure nationale et on les disques on liste les grandes catégories, on prévoit un mécanisme d'association de la réindustrialisation, ne peut pas être un sujet. Qu'on met sous le tapis. Il est nécessaire pour des questions de transition écologique. Il est nécessaire pour des questions de souveraineté. Mais je ne vois pas comment on peut, malgré la qualité du travail de cette assemblée, poser des principes on va ajouter des gigafactories à des éléments sur lesquels on a des difficultés à définir et la proposition qui vous est faite dans le cadre de l'amendement que je vous présente ça c'est qu'il y aura dans le PJ l'industrie verte. Avec le temps qui se poursuit en particulier avec les commissions économiques des deux chambres, la définition de ces grands projets d'envergure nationale à caractère économique qui viendrait dans le cadre de la discussion parlementaire s'ajouter mais qui permettrait d'associer les commissions. Qui ont déjà commencé à travailler avec Bruno Lemaire sur une partie de ses sujets et de ces questions, donc on botte pas en touche mais on a une procédure pour les intégrer parce que sinon la porte de qui économique peut être relativement large enfin une fois qu'on a dit qu'on avait ses grands projets d'envergure nationale avait ses projets économiques qui, trouver une place dans le pays à l'industrie verte. La question qui reste et. Quel comptés à part pour ses grands projets d'envergure nationale. Et la position qui est celle du gouvernement et de dire. On les compte dans une enveloppe nationale mais il ne disparaissent pas de la trajectoire d'artificialisation. Parce que ce sont bien des hectares qui à un moment ou un autre participent à l'artificialisation. Et donc on assume une péréquation par région. En l'état actuel du droit, ce qui n'est pas supportable. C'est qu'on a des territoires qui se retrouveraient privés d'une très grande part de leur capacité à agir à cause du poids des infrastructures nationales. C'est particulièrement vrai pour les de France qui est la région qui est la plus touchée, mais il y aurait une sorte de double peine pour des territoires qui ont attendu pendant longtemps des infrastructures de désenclavement. Parce que non seulement. Elles n'ont pas bénéficié par le passé de ces infrastructures, je pense à l'Occitanie. Mais en plus. On viendrait leur expliquer qu'elle doit faire moins tout en intégrant ses infrastructures là où ceux qui ont eu les infrastructures aurait le droit à la moitié de ses infrastructures dans la trajectoire sans avoir besoin de les reconstruire d'où. Ce comté à part mais qui ne disparaît pas deux l'artificialisation parce qu'à la fin ça partie bien au recul des Terres agricoles et des espaces naturels dont on a besoin pour préserver la biodiversité. Voilà l'amendement 3 points. Hein comptés à part qui ne fait pas disparaître l'artificialisation une liste des grands projets d'envergure nationale qui permet une discussion et une procédure spécifique avec les commissions économiques de l'Assemblée et du Sénat pour la partie industrielle. Merci monsieur le ministre et le 2ème amendement. Est présenté par Monsieur Johanet le 109 rectifié. Merci monsieur le président. j'entends bien ses propositions pour le compte et à part. Cet amendement vise lui a ajouté à la liste des projets non comptabilisé les projets qui représentent un intérêt écologique, puisque vous connaissez Monsieur le Ministre, sur l'ensemble de ces bancs notre fibre écologique. En particulier l'ensemble des projets d'infrastructures qui concourent à la transition écologique. En effet, la mise en oeuvre du zéro artificialisation nette dans les territoires ne doit pas entrer en opposition avec d'autres objectifs poursuivis en matière de transition écologique, en particulier la décarbonation des activités humaines, l'efficacité énergétique. L'économie de ressources ou l'adaptation des territoires en charge au changement climatique. Par ailleurs, dans d'autres domaines comme. La gestion et le stockage des déchets. les objectifs ambitieux que nous nous sommes donnés en la matière nécessite la multiplication de plateforme par exemple de recyclage qui peuvent là aussi nécessité du foncier au regard de ce qui précède le présente le présent amendement pardon propose d'exclure les projets d'infrastructure qui participe à la transition écologique et énergétique de toute comptabilité afin d'encourager leur réalisation rapide de concilier ainsi l'ensemble des efforts qui doivent être menées simultanément en matière de transition écologique. un amendement peut-être quelque peu ambitieux mais qui méritait d'être portées au débat. Merci monsieur le rapporteur. Sur ces deux amendements.

La gouvernance et bien entendu important mais le mais celui le sujet des grands projets c'est. Plus que. Fondamental. Déjà le fait que les décrets revienne sur la loi a participé à créer un malaise. Dès le, dès Ensuite cette impression. Alors c'est toujours pareil. L'impression le ressenti que l'État définisse seul les grands projets. N'a pas aidé l'Assemblée. Dans le cadre de ses travaux. Et puis cette impression aussi que l'État s'exonérer lui-même de ce qu'il impose aux collectivités locales, donc ça se tiendrait pas aux mêmes obligations de sobriété foncière dans le cas de sa trajectoire. Et puis quelques réponses à et là qui ressemblerait des arguties juridiques ou. Ou un État qui chercherait à devenir une fiction juridique. Et on le voit un peu quand vous dites, Monsieur le Ministre, que les hectares ne disparaissent pas. Voilà alors nous avons donc bien de problèmes devant nous au moins c'est définir les grands projets. Merci de préciser qu'il a un projet de loi à venir et qui va nous aider en ce sens, et ensuite il y a le comté à part. Voilà cette assemblée, me semble-t-il, ça s'est traduit dans cette commission spéciale. Souhaite par la conférence régionale donner des avis sur des grands projets proposent des critères qui nous paraissent Simple sur qu'est-ce que des grands projets. Et ensuite, souhaite un vrai comptés à part dans une création d'un compte national pour que l'État s'applique à lui-même, c'est qu'il applique aux autres et participe à l'effort national de réduction de l'artificialisation. Des sols. Donc c'est comme ça que la, la commission a travaillé à ce stade là. Bien entendu et des marges de progrès pour tout le monde. Mais c'est pour cette raison que c'est à mon avis sera défavorable. monsieur le rapporteur. Donc, avis défavorable. De la commission sur ces amendements et j'imagine, avis défavorable du gouvernement sur le 2ème amendement puisqu'il en propose en lui-même donc. Donc j'ai de demandes d'intervention Madame brûlant. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues j'ai j'ai bien écouté la démarche que vous proposez, Monsieur le Ministre, j'y vois plusieurs écueils d'abord. J'ai en mémoire que lorsqu'on a examiné ici le projet de loi d'accélération du nucléaire. Il a été question d'un certain nombre de lien, évidemment avec Cezanne et on nous a dit en gros, ça pourrait être discuté au moment Dusan en ce moment même, alors que le texte accélération du nucléaire est à l'Assemblée, on dit à nos collègues députés. Lausanne, ils sont en train d'en parler au Sénat. Attendez votre tour ça reviendra et puis là vous nous dites qu'il va y avoir un autre texte. Industrie verte. Qui va prendre en compte d'autres choses, c'est quand même un peu compliqué de ne pas examiner les projets dans leur globalité, c'est un peu sans faire de provocation de bas étage, comme quand on nous dit il y aura une loi travail après la loi, retraite, ne vous inquiétez pas, le meilleur est à venir. mais au-delà des suspicions ou des doutes qu'on peut émettre les uns et les autres, je pense que cette logique ne permet pas de prendre en compte la globalité des choses, exemple dans mon département, il est question en tout cas je le souhaite, à titre personnel et même un peu au-delà d'accueillir 2 réacteurs EPR. Mais accueillir les réacteurs EPR, ça va avoir une implication sur Lausanne qui serait pris en compte dans les grands projets que vous venez d'évoquer, mais ça a aussi un impact que parce qu'il va falloir accueillir 7 à 8000 salariés et que à ce titre-là il faut construire des logements, il faut faire venir des médecins, il faut créer des formations etc etc qui roi aussi un impact sur Lausanne or. Pour l'instant, nous ne prenons pas je trouve en compte la globalité de ça, on prend l'emprise foncière des 2 réacteurs. Et on ne prend pas en compte la globalité en termes d'aménagement que le territoire au sens large va devoir mettre en place et je trouve que c'est regrettable pour notre réflexion et qui auraient besoin d'assurer un peu plus de cohérence. Merci. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Effectivement cet article et les propositions qui sont faites par la Commission et l'amendement du gouvernement sont aussi un des points. de de ce projet et et si je comprend bien la logique que l'on partage de mutualisation, le fait de remonter. Les projets nationaux, je ne parle pas de la manière dont ils seront définis qui qui est aussi un sujet. Semble pouvoir être assez largement partagé la question ensuite c'est comment on les faire redescendre puisqu'en fait c'est ça votre intention. Et là, je voulais juste. Faire part de de 2 observations, la première c'est que certes les territoires qui ont la chance d'avoir des projets d'intérêt national, ne peuvent pas être pénalisés et, et ne peuvent pas. Faire valoir la totalité de leurs quotas de 2 pour les accueillir. Mais ils ont aussi la chance je lisais de les accueillir donc de d'avoir un, un certain développement économique qui est induit et des créations d'emplois de l'activité. Ce que les territoires qui n'accueillent pas ces projets nationaux. Non pas alors que il serait contributeur au prorata si on devait faire redescendre. Une partie de ses projets nationaux sur l'ensemble des des territoires. Donc moi je souscris plutôt à la proposition de la Commission spéciale qui est de dire il faut qu'il y a un comptés à part pour ses projets nationaux parce qu'effectivement ils ne peuvent pas peser sur les seules régions qui sont concernées, mais ils ne peuvent pas non plus venir imputer les quotas ou les capacités de territoire qui n'ont pas la chance d'accueillir des projets nationaux et je vais pas plus loin pour me prononcer sur les sur les projets sur Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Permettez-moi d'illustrer je dirais ce que vous avez expliqué comme. Sélection j'allais dire des projets si vous avez cité, Les Hauts de France. Je suis sénateur de la Somme. Aujourd'hui si les grands projets qui sont, je vais vous les citer bien sûr le canal Seine-Nord Europe 2200 hectares le port de Dunkerque 3000 hectares les parkings du Brexit 100 hectares le passage 2 fois 2 voies de la RN 2 Laon Avesnes sur Helpe. Sans hectares si on compare par rapport à la consommation des 10 dernières années et qu'on fait le prorata pour le grand Amiénois c'est-à-dire la région d'Amiens, très attractive en cette période, il nous reste 15 hectares par an. À consommer. Sachant déjà que pour l'année 2023. Amiens attends 50 hectares pour une, une entreprise qui peut créer des panneaux photovoltaïques, 30, 20 à 30 hectares pour une usine très novatrice pour des créations de pile à sodium d'une là qui sont s'appelle Tihama. Vous voyez donc bien que l'illustration. De ce cas et tout à fait. Pas Monique de la difficulté que vont avoir les territoires, si on exclut pas un certain nombre de projets. Deux européens, mais également certains régionaux.

Ça va consommer du français. Si vous faites de la mutualisation, vous allez demander à toutes les régions de participer à fournir finalement une part de foncier disponible. Carlos Saura les retombées, sachant que ces régions vont perdre leur recette puisque c'était du foncier disponible sur lequel ils n'auront pas les impôts. Et qu'alors les autres régions qui auront sur leur territoire les centrales nucléaires pour prendre cet exemple auront des recettes extrêmement importante et j'ai cité par exemple l'exemple de Paluel ou si on compare les revenus par habitant, c'est de l'ordre de 7000 euros par habitant, et pour les communes qui sont de strates et identique. Ces 500 euros. Comprenez que de mutualiser du français sur lequel on perd des recettes va poser énormément de problèmes pour les territoires. Merci monsieur Corbizet. ce qui risque à avoir aussi un conflit d'intérêts économiques et financiers. C'est-à-dire que vous avez un secteur que envie de s'inscrire sur une liste nationale, le projet d'intérêt national et puis elle va être retenue pour des raisons stratégiques, pourquoi pas politique. Puis après, le gouvernement se retournera sur les collectives locales, régions, départements impression ben nous on l'a retenue au niveau national, maintenant vous avez co-, financer les projets aucun autre côté est-ce que cette fameuse conférence régionale a directement Dusan puisqu'aussi c'est les sur les régions que la compétence développement économique parce qu'à un moment donné il peut pas y avoir un choix de projets d'intérêt national qui transitent par les conseils régionaux. Merci Monsieur Dantec. monsieur le président. Moi, on est sur un, un débat important même si j'ai bien entendu. L'alerte de Madame l'état. Se trouve que le l'amendement du gouvernement va quand même dans le bon sens d'éclaircir la position du du gouvernement. Il me semble quand même qu'on a besoin d'un dialogue avec les régions à l'échelle nationale. Je pense que. Je crois qu'au niveau il faut et c'est c'est pas contradictoire avec ce qui a été proposé que que les régions. Soient consultés au niveau national sur les projets qui rentre. Effectivement dans ce conte nationale. Puisque derrière il sera ré-imputés. Aux différentes régions, ce qui est certain et c'est un point sur lequel on est tout à fait d'accord. Avec Monsieur le Ministre, c'est que si on n'a rien pu de porc. On va essayer de tout mettre dans le. National, quand on va, on va avoir une liste permanente. On va essayer et on trouvera toujours une part d'impact national de tel ou tel projet, donc on n'en sortira pas. Et je pense que effectivement appartement il y a une imputation sur les régions qu'il a un dialogue, il faut probablement inventer un lieu de dialogue, les régions elles-mêmes mettront le holà sur le fait remonter trop de choses sur le, sur le compte national et l'équilibre se fera peut-être un moment de tâtonnements et de tension mais ça devrait fonctionner. Voilà Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure par ma collègue communiste. D'après les les. Nos dernières infos de de sources scientifique très sûr entre les Lions. On ne peut pas mais les centrales nucléaires parce que l'eau des rivières sera trop chaude et les endroits où il y a un risque de submersion marine je on s'est vraiment de source sûre que tout le monde travaille actuellement sur un projet de localisation unique de tous les réacteurs EPR sur un seul site, un peu comme des Lego avec des réacteurs empilés les uns sur les autres, donc l'emprise au sol sera au final négligeable. Madame Cukierman. Les dernières phrases pardon de de notre collègue Laurent Somon puisque nous avions envisagé de déposer un amendement pour demander un simple rapport. Sur la question de la fiscalité locale. Il a été déclaré Heroes. Solvable et pourtant si je reprends les derniers propos et on le voit bien et on va le revoir, je n'en doute pas, à travers d'autres débats sur ce texte, il y a réellement un rapport entre la fiscalité locale. Et l'enjeu Dusan. Et il est à plusieurs niveaux. La question bien évidemment. Du devenir d'une recette qui aujourd'hui et la taxe foncière. On dirait bon l'avantage c'est que comme il y a plus la taxe d'habitation ce débat là est réglé mais il reste quand même encore la taxe foncière. La vraie question, si on va jusqu'au bout de la démarche, je ne dis pas que c'est ce qui est affirmé. Mais si à un moment donné on arrête de construire. On on ne gagne on gagnera de moins en moins d'habitants dans un certain nombre de communes. Or aujourd'hui on sait que l'apport de la DGF, on sait, oh combien les collègues élus sont en panique au moment du recensement. Pour savoir à quel niveau. L'on va l'être. certains demandent même parfois. Des. Recalcule auprès de l'Insee, parce que cela a des incidences effectivement sur la DGF et donc sur la capacité de la commune à pouvoir investir après donc on sent bien qu'on a finalement une fiscalité locale. Hérité de de de de de de d'année sans âme. Et si on ne la repense pas au sens plus large. Le Zamme de toutes les façons ne marchera pas. Donc moi, Monsieur le Ministre, je pose également cette question à travers tous ces, ces questions de grands projets. Comment est-ce qu'à un moment donné, cela a un impact sur la fiscalité locale. Comment vous l'anticipez très certainement dans une prochaine loi décidément on va avoir beaucoup de prochaine loi mais avec grand plaisir. Merci monsieur Boyer. Oui, merci Monsieur le président. Je crois que avec ce sujet là, on touche vraiment au coeur. De la proposition de loi qui est faite aujourd'hui. Lors des différentes auditions qu'on a pu avoir. Dans. Dans les différentes réunions, on s'est aperçu. Et lorsqu'on a auditionné des responsables de régions en particulier. Que lorsqu'il sortait l'ensemble des projets qu'ils avaient sur leur territoire. Il restait quelques hectares en peau de chagrin. Pour le reste des communes. Dès qui vous qui pouvaient être concernés. Donc si on ne sort pas. Des surfaces qui sont. Prises sur des projets d'envergure nationale, voire des gros projets régionaux. Si on est 100, pas en termes de surface. Il ne va rester pratiquement très peu de choses en termes de surface organisé pour les communes qui sont sur, c'est que ces ces périmètres que sur sur des métropoles, voire même sur des communes rurales. Donc on est vraiment au coeur du sujet et si. On ne résout pas ce problème-là. On va au devant. De. De surface qui seront pratiquement inexistante pour les collectivités. Donc. En dehors du problème financier qui est posée par mon collègue tout à l'heure qui a été posé. Le problème de la, des surfaces elles-mêmes il vrai cruellement posée aujourd'hui sur cet aspect-là. Donc Monsieur le Ministre. Il faut vraiment qu'on est votre position. Et votre sentiment par rapport à ça parce que si si. Si on n'a pas une assurance dessus, enfin je veux dire que on on est vraiment sur. Une une une partie qui est déjà joué et qui est terminée pour l'ensemble des des Si Monsieur le Président. La le compte part des grands projets. Je crois qu'on on tombera d'accord là-dessus. C'est c'est c'est une évidence qu'on est obligé de, de passer par là. En revanche la réputation, permettez-moi de m'interroger sur. La façon dont elle va pouvoir être réalisée. À part ce qui porte et qui ont, qui ont des des projets en nombre et ça été rappelé l'exemple de Hauts-de-France c'est assez parlant leur en ce moment-là la rappeler. Mais il y a d'autres régions aujourd'hui qui ont beaucoup moins de projets, voire pas de projet. Carrément pas de projet. Comment va-t-on re-amputé. C'est c'est compter à part si on doit le faire. Entre ceux qui ont déjà presque tous eu hein et qui effectivement. Ont Ont moins de besoins que les autres et qui en plus vous l'avez rappelé auront des droits parce qu'ils ont consommé. Sur la période passée. Et ceux qui n'ont pas grand chose. En terme d'équipements désenclavement ou autres et j'en sais quelque chose hein quand on attend depuis longtemps des désenclavement ferroviaire routier en Haute-Vienne par exemple. on est doublement pénalisés. Ça va être très compliqué de discuter de de critères de réputation donc permettez-moi sur ce sujet de, d'avoir de sérieuses réserves sur. L'équité territoriale qui pourraient en résulter. Merci madame Préville.

Moi je vous parle d'un territoire. Le nord du Lot où on peut considérer qu'on est les oubliés du ferroviaire. Mais, mais vraiment à la ligne Polt Paris-Orléans Limoges Toulouse est déclassé à partir de Brive. C'est-à-dire qu'entre Brive et Cahors. Moins de trains moins de desserte. Et nous sommes bien évidemment très loin de Montauban qui sera la future gare d'accès à la ligne LGV et donc concrètement dans ce que vous nous présentez ses objectifs qui doivent être déclinées. Territorialement vont nous impacter nous alors que et Christian l'a dit, il n'y a pas d'équité territoriale, au niveau du fait du ferroviaire dans notre pays et particulièrement sur quelques petits territoires isolés comme le mien. Nous on sera loin, on n'ira jamais à Montauban prend la LGV et puis on est obligé d'aller à Brive avec le peu dessertes qu'on a dans le Lot avec très peu de trains et vous le savez fort bien sur la ligne Polt

On est vraiment. Voilà je c'est c'est c'est quasiment impossible pour nous d'envisager ça et comme le dit Christian c'est la double peine. On n'a pas. Le le service et en plus on va être impactée sur un territoire très rural, 174.000 habitants dans le Lot et donc très peu de d'offre de mobilité. Monsieur Delcros. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre. On voit bien à travers ce débat on touche un point sensible qu'on retrouve. Sans doute d'ailleurs tout au long de de l'examen de ce texte qui est la question de l'équilibre dans le traitement des territoires. Certains collègues ont parlé de double peine, et caetera. Il faut qu'on fasse des ou d'équité territoriale, il faut qu'on soit très vigilant. Et on ne peut pas. Pénaliser 2 fois doublement en quelque sorte. Les départements qui ne bénéficient pas des infrastructures, ce qui bénéficient, pas d'infrastructures non pas les emplois qui accompagne ces infrastructures, non pas les richesses souvent qui les accompagnent et et devraient réduire leurs droits à construire en raison des infrastructures qui sont réalisées ailleurs je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant là-dessus je pense ça va être d'ailleurs une ligne dans l'examen de ce texte de toujours veiller à. Un traitement équilibré des territoires et en tous les cas ne jamais appliqué. Le régime de la double peine. Voilà c'est, je pense que. C'est la raison pour laquelle il me semble que ça n'est sans doute pas la bonne solution que de venir réintégrer d'accord pour une enveloppe nationale mais devenir réintégrer. Ces ces superficie de l'enveloppe nationale dans l'ensemble des territoires de France. Oui, merci Monsieur le Président. Ce le rapporteur sur le midi, chers collègues. Je voudrais prendre un exemple très concret, le gouvernement aujourd'hui et au niveau du Sénat, nous avons voté ce texte. Sur la relance du nucléaire, ça fait longtemps que le Sénat considère qu'il est absolument essentiel d'avoir un plan ambitieux de production énergétique décarboné horizon 2050 et le nucléaire en fait partie. je j'évoque ce. Ce point là Monsieur le Ministre, c'est que le Sénat qui a examiné en première lecture avant l'assemblée parce que l'Assemblée seulement en train le d'en débattre

Considérant que c'est un enjeu national, ce qui est vrai, une centrale. L'ambition n'est pas propre au territoire mais bien d'alimentation d'envergure nationale. je j'interviens cet instant Monsieur le Ministre, c'est parce que les choses sont en train de bouger au niveau communautaire et la Commission vient d'exclure. De sa reconnaissance de toute la liste qui était donc il y a toutes les énergies, sauf qu'on vient de sortir le nucléaire à nouveau on ne refait le coup de la taxonomie qu'on a connu sur lequel on a dû combattre et où aujourd'hui on sort le nucléaire. De la considération des. Du zéro. Émission nette. Et si je vous pose la question Monsieur le Ministre, c'est qu'effectivement on voit bien que la France est à nouveau interpellé sur ses choix stratégiques et comment nous allons pouvoir effectivement prendre en considération cet aspect des choses au niveau de nos territoires sur l'enjeu énergétique et le quelque part la non pérennisation de territoire par rapport à l'implantation des sites des futures centrales. Merci, monsieur le Président, j'ai entendu. Madame la présidente, et donc. Je vais gagner le le temps de parole sur la présentation de la manne demain les je crois de. Mais je voudrais réagir en disant que, effectivement, ces grands projets. À mon sens il faut les mutualiser. Ses projets d'nationaux mais c'est quoi un projet d'intérêt national. Je vais être avec un peu de facilité, Monsieur le Ministre. Vous vous mettez les établissements pénitentiaires que ne résiste pas dans cet hémicycle Victor Hugo à ce que je veux dire. De rappeler que quand on ouvre une école on ferme une prison. Les écoles ne sont pas convaincus. Que je sache c'est l'éducation nationale. Donc quand on ouvre une école quand on ouvre un collège quand on ouvre de l'huissier. Un projet d'intérêt national. Je rappelle que les gendarmes vivent dans des conditions souvent dramatiques dans des logements insalubres d'. C'est C'est la gendarmerie nationale. Si on ouvre une caserne de gendarmes d'ailleurs le chef lieu de canton. C'est un projet national et ça doit être mutualisé. Donc c'est très compliqué, mais moi je crois que lorsqu'on agit pour l'intérêt public, on est dans un projet d'intérêt national et que ça doit être décompté du territoire parce que les territoires qui ont moins nectar. Quand ils devront construire un collège il ne restera 0 m2. C'est-à-dire que nos rien faire un entre. Et pourtant les feront en train de construire pour l'éducation nationale, donc c'est un sujet très complexe. Madame Lienemann. Moi je crois qu'une des difficultés que nous avons c'est que nous avons qu'une estimation un peu planifié. De quels vont être non seulement les projets nationaux. la réindustrialisation du pays. Quand on va pas réindustrialiser qu'avec des grands deux gigafactories. On va aussi essayer de développer des ETI. La plupart de ces ETI ne vont pas s'installer dans les centre-, ville où les zones hyper urbanisée. Ici ou là on trouvera des friches. Mais si on veut réindustrialiser le pays, faut au moins une certaine estimation de combien ça va avoir d'impact sur l'artificialisation des sols. Et on est en train de faire comme si. Toutes nos ambitions. Allez pouvoir rentrer dans une bouteille. Même s'il y a 3 litres d'eau et que la bouteille ne fait qu'un litre. Donc moi je suis évidemment favorable Lausanne mais avec un principe de lucidité, de vérité. Quelle est l'estimation réelle qu'on peut faire pour les 10 ans à venir. Nécessaires pour réindustrialiser le pays réaliser les grands projets, voir si tout sont indispensables. Ça c'est, c'est encore autre chose. Et qu'est-ce qui reste ensuite à l'aménagement plus entre guillemets micro-locales, régionales ou locales. Et on fait comme si, une fois qu'on va avoir déclaré la la loi. On va pouvoir résoudre ces problèmes. Et ben il y aura 2 solutions, soit on va dire non à des implantations d'activités économiques d'avenir soit on va déroger encore Uzan et je le dis tout Net, j'ai quand même l'intime conviction qu'en dépit du travail de qualité, fait par notre commission qui limite la casse. On y va à l'aveugle et ça n'est pas sérieux. La plupart des autres pays ne se fixe pas des contraintes aussi borné avant d'avoir étudié quelle était l'ampleur des mutations qui se présenter devant eux pour les 10 années à venir. L'âme Espagnac. Oui je vais me si Monsieur le Président, je vais rebondir sur ce que vient de dire Marie-Noëlle Lienemann je sens qu'on a trouvé du travail pour le haut commissaire au Plan, la sénatrice des Pyrénées-Atlantiques je suis. Est ravi d'avoir trouvé une nouvelle mission à monsieur Bayrou. En plus de ses fonctions précédentes blague à part, Monsieur le Président, veuillez m'excuser, je voulais juste dire à Monsieur le Ministre rajouter peut être un élément par rapport à l'intervention de ma collègue Angel. Préville sur la double peine qu'elle évoquait pour pour son territoire, Monsieur le Ministre. Et pour vous dire qu'en fait ce n'est pas une double peine puisque c'est une triple peine, en fait elle a oublié un élément en plus de l'impact Dusan et en tout cas de de la compensation sur Lausanne donc sur le, les grands projets et notamment sur les transports qu'elle n'aura pas, il se trouve qu'elle va payer en plus enfin toutes les communes. Aux alentours qui vont être impactés par Lausanne vont payer en plus l'impôt LGV

de transport comme cela a été dit, donc je tiens à vraiment à a insisté sur le fait de faire très attention en tout cas sur l'impact que les communes qu'on sous-estime peut-être mais, potentiellement, vous voyez bien, même il y a quelques semaines ou vieux vous nous votions ici un impôt sur sur la LGV, qui va encore là là aussi impacté les communes dans leur ensemble, donc je pense qu'il avait prises en compte général à à observer de près. Bien merci avant qu'on passe au vote je redonne la parole à Monsieur le Ministre. Mes chers collègues d'abord de quoi on parle. En nombre d'hectares. Si j'additionne les grands projets d'envergure nationale qui font partie de la liste potentielle qui vous est soumise. On est avec un biais optimiste qui considérait que tous les projets sont réalisés en 2031. Cette Nord Europe LGV et compagnie, sur l'équivalent de 10% de l'enveloppe nationale. Dit autrement, en terme de péréquation. Là aujourd'hui, Les Hauts de France ont 60% de grands projets d'envergure nationale dans leur enveloppe globale ce qui a été dit pour la somme est exact. On serait sur un schéma dans lequel on serait à 10% de moins pour chaque région de manière à tenir compte du partage de tous ces grands projets d'envergure nationale. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, je me permets de dire à la sénatrice Préville a une partie d'entre vous. Faisons attention quand même à ne pas nous couper les cheveux en 4. À partir du moment où vous fixez une maille régionale. Et où il y a des projets qui, à l'intérieur de la région ne sont pas dans chaque commune de chaque département par définition il y a un partage de l'enveloppe foncière. Mais c'est comme si demain on considérait qu'à l'intérieur d'une communauté de commune, il n'est pas normal qu'une ligne de transport en commun qui ne traverse pas Maru dans ma commune. Participe. D'un financement qui soit intercommunal alors que j'en bénéficie pas. Quelle est la maille jusqu'à laquelle on descend jusqu'où on va pour le fait de les considérer ce qui relève des uns et des autres, parce que si vous commencez à le faire. Le sujet c'est pas seulement infrastructures. C'est l'usage. Est-ce que le fait d'avoir une ligne de rails. Participent à la décarbonation, est-ce que c'est le fait d'avoir des trains dessus à quelle fréquence. Et à ce qui est ce moment-là il faut coefficient T une partie du dispositif, en fonction de la réalité du service. Donc ce que je veux vous dire. C'est que plus on va entrer dans un degré de complexité. Plus le risque qu'à la fin, on trouve des raisons de ne pas faire deviendra grand. Hein. Tout ce dont on discute dans cet art. Si ce n'est pas un problème de décret, c'est un problème de loi. Si on en reste là si on garde le texte de la loi climat et résilience, tout ce que vous avez décrit comme étant un problème s'appliquera tout ce qui est proposé, que ce soit par la commission ou par le gouvernement c'est pour corriger. Une loi qui n'a pas intégré cette dimension. Il y a des choses qui sont extrêmement simple. Une centrale nucléaire. Une prison ça c'est simple. À partir du moment où on a un arrêté. Une DUP nationale. On est dans la catégorie grand projet d'envergure nationale et on a une catégorie qui est compliqué parce que des projets industriels peuvent avoir un intérêt mais comme ils sont portés par le privé. La porte d'entrée peut pas être la même. D'où. Le pays à l'industrie verte qui va permettre d'essayer de lister une partie tout ça parce que ça nécessite un travail je vous le dis comme je le pense qu'il doit se faire avec le ministère de l'économie et avec les commissions concernées pour être capable d'aller préciser les éléments. Une fois qu'on a dit ça. Je le pense sincèrement. Les enveloppes foncière dont nous disposons. Les friches qui existent dans notre pays rendent largement compatible ses ambitions pour les 10 ans qui viennent avec ce que nous sommes en train de dire. L'argument que les autres. Font serait tête baissée, n'est pas exact. L'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suisse j'ai énuméré la liste de ceux qui sont sur du zéro artificialisation nette avec des dates qui sont comparables aux nôtres. 2ème point. Nous avons aussi à l'intérieur de tout ça des marges. Encore une fois quand on se souvient que la moitié de la consommation foncière. Ça a été pour accueillir des lotissements avec moins de 8 logements à l'hectare, ça montre qu'on a quand même on part pas d'une situation on a plus un mètre carré disponible parce que tout serait danse et on a dans le schéma dans les corrections vous proposez dans les allers-retours qui sont imaginer des dispositifs qui nous permettent d'avancer et donc j'assume. La nécessité d'une réindustrialisation, avec un dispositif Haddock une liste de grands projets d'envergure nationale qui prévoient toutes les consultations des élus locaux pour être certain qu'on les reprenne à notre compte. Et enfin, et c'est là-dessus que je terminerais on vous entendant ce soir je suis plein d'optimisme. Pas sur l'issue du débat législatif ça par définition on trouve un chemin. Parce que je ne vois que des gens qui veulent réindustrialiser qui veulent lotir qui veulent accueillir des projets industriels qui veulent accueillir des habitants. Je tiens à vous dire qu'on a en parallèle. En parallèle. Un recul des signatures de permis de construire. Comme on en a rarement connu et qui n'est pas que le fait de la montée des taux d'intérêt d'un côté et du coup de l'immobilier, de l'autre. On a. Une montée. On a une montée de beaucoup de riverains qui ne veulent pas de voisin. On a. Allez dans les communes discuter voyez la difficulté à faire en sorte d'aller valider un projet. D'urbanisme ou tout simplement a permis de construire dans une rue aujourd'hui. Aller mesurer la manière dont les riverains accueillent des projets de réindustrialisation. Avec les inquiétudes sur les nuisances économiques qui sont liés à ça. Et entendez la réaction d'une partie de nos collègues élus locaux qui ne se pressent pas pour accueillir des promoteurs et pour favoriser des projets donc au-delà des débats. Que nous portons. C'est étonnant de regarder comment entre la part des DMTO, la part de la taxe foncière. La réalité, précisément de. Ses impôts et de leur dynamique considéré qu'il n'y a pas de produit fiscal. D'abord ce serait être un peu court, et ce serait ensuite supposer que le seul intérêt d'un élu n'est pas d'abord de regarder comment il répond au service et il permet de faire progresser la population mais comment il augmente les recettes de sa commune. Ça ne correspond pas à mon expérience personnelle donc mesdames et messieurs les sénateurs. La proposition qui vous est proposé. Ce soir, elle a le mérite de définir une porte qui corrige la loi telle qu'elle existe. De proposer un mécanisme d'association sur la partie économique dont vous conviendrez qu'il qu'il faut qu'on la dimension correctement parce que si tout ce qui est privé n'est plus de l'artificialisation on a un autre souci. Et qui propose à la fin en pourcentage. Un volume de 10% qui n'est pas incompatible avec la poursuite des autres objectifs que nous poursuivons par ailleurs. Bien, merci Monsieur le Ministre, nous allons passer au vote, sur les deux amendements monsieur. Oui, éclairé par tout ce qui vient d'être dit et considérant que mon amendement était peut être. C'est des peut-être une dimension beaucoup trop ambitieuse en matière écologique. Je vais le retirer. Bien, donc il nous reste l'amendement du gouvernement dans les deux amendements que vient de en défendre à nouveau. Monsieur le. Le ministre avec un avis défavorable de la commission. Donc, je le soumets aux voix qui est pour l'amendement 181. Qui est contre. Il a. Qui s'abstient. N'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 24 rectifié monsieur Sautarel. est très faible, il y avait un rapport. Qui s'intitulé futurs énergétiques 2050 de RTE qui le démontrer concernant les installations photovoltaïques. Et donc cet amendement pour pour aller vite propose une pérennisation au-delà de 2031 de la présomption de non-artificialisation des sols pour les installations de production d'énergie photovoltaïque qui n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol et applicable à cette présomption aux installations agree photovoltaïque au sens de l'article L. 314 36 du code de l'énergie. Je veux juste profiter d'un petit temps de parole qui m'est offert à cet instant pour défendre un amendement ou du moins rappeler un amendement qui a été déclarée irrecevable au titre de l'article 45. Ce que je comprends tout à fait mais qui me semble centrale quand même dans le sujet que l'on traite et sur lequel il conviendra de revenir. C'est la place le rôle des des Cdpenaf parce qu'on parle beaucoup ici de l'orientation. On parle beaucoup de la stratégie, on parle de la planification mais ensuite dans la mise en oeuvre et dans les décisions, la place des Cdpenaf est absolument essentiel. On a beaucoup évoqué. les libertés locales et la place des élus dans les instances et donc mon amendement visait à renforcer la place des élus locaux dans les Cdpenaf de façon à ce qu'il soit vraiment le représentant de l'intérêt général dans les décisions qui soient prises et donc je pense que ce point-là devra être revue. Parce que c'est un élément essentiel dans le pilotage de l'urbanisme et de l'aménagement de nos territoires. Je vous remercie. Merci. Avis du rapporteur sur l'amendement 24 rectifié. Oui, monsieur le président, mes j'ai mes chers collègues, que c'est effectivement un sujet que nous avons traités dans la dans la commission. Mais qui considère que en

Identique. D'abord parce que dans le cadre de la loi sur le l'accélération des énergies renouvelables. On précise bien qu'on sort de l'agrivoltaïsme. On sort aussi de l'agrivoltaïsme une partie des projets à condition qu'il y ait des conditions de hauteur pour que la biodiversité puisse se reproduire en dessous d'espacement et qui je pense ont plus fait l'objet de débats. c'est la raison pour laquelle où il est satisfait sous cet angle-là, ou si on généralise il pose une difficulté parce qu'il nous conduirait à devoir revoir la typologie de ce qu'on a classés en agri-voltaïque ou en photovoltaïque.

Oui, donc très rapidement hein. On revient sur ma ma prise de parole précédente hein. C'est pour. Affecter à l'enveloppe nationale tout ce qui est. Bâtiments. Publics qui sont. Dépendants des missions régaliennes de l'État. J'ai les, les écoles, les collèges les gendarmeries. Il ne concerne pas le territoire sur lequel ils ont construit la commune, faire les gens construit et donc ils doivent être dans l'enveloppe nationale. Même s'ils n'ont pas une grande superficie.

Et moi je me dis que pour avoir un espace agricole il faut 2 choses. Il faut du terrain agricole. Et il faut un agriculteur. Pour l'entretenir. Parce que s'il n'y a pas d'agriculteurs. Il n'y a pas de terrains agricoles. Alors l'agriculteur. Vous savez tous plus ou moins et est mal en point. Alors on a des j'études, des enquêtes. On a même des rapports sénatoriaux. Qu'il nous faut inverser leurs larmes sur le chouchou des agriculteurs. Mais il y a aussi la difficulté de transmission, avait des bâtiments, souvent vétustes. Et donc moi je dis que si on veut sauver les Terres agricoles. Il ne faut pas compter les bâtiments d'exploitation parce que le bâtiment d'abstention. C'est pas une artificialisation. C'est la nécessité. Pour avoir des Terres agricoles parce que si on n'a pas de bâtiments d'exploitation. On n'a pas l'agriculteur et si on n'a pas d'agriculteurs, on n'a pas de Terres agricoles, le bac, il va l'exploitation c'est une préservation de l'environnement. Le bâtiment agricole. Bien merci donc ont été présentés le 62 rectifié et le 63 rectifier le 41 rectifié le président Longeau. Oui, merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. cet amendement il vise à reconnaître. L'intérêt écologique de certains projets et à ouvrir le Champ à des exonérations de comptage. Dusan pour ces derniers, en matière d'économie et de ressources. La loi La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a fixé des objectifs ambitieux en matière de gestion et de stockage des déchets. Son exécution implique la multiplication de pare-feu de plateforme de recyclage notamment pour un effet important, celui de lutter contres les décharges sauvages et préserver les sols le autre d'amendement proposant enfin des. Les projets d'infrastructure qui participe à la transition écologique et énergétique. Je vous remercie.

Je ne souhaite pas forcément battre le record de notre collègue Raymonde Poncet Monge pour laquelle nous avons néanmoins à cet instant une pensée puisque ce sont des sujets écologiques qui s'applique. Et donc considérer que l'amendement est défendu.

Merci Monsieur Monsieur Nice, simplement pour dire d'abord qu'il est défendu mais j'aimerais que Monsieur Miss nous précise bien que les gendarmerie nationale Robert bien impôt national parce qu'on a lu dans la nomenclature qui avait bien les centres pénitenciers pas les gendarmerie nationale et 2ème point pour revenir à ce que dit mon collègue Billac. Attention aussi au fait. Lorsqu'on parle d'une terre agricole qu'on parle d'un agriculteur, qu'on fasse attention aussi que ce soit un vrai agriculteur et non pas un ancien agriculteur qui soit devenu ça ça ouvrier d'une grande entreprise de BTP. Ou d'assurance hein et qui se construisent des grands bâtiments ou déchets avec des architectes de renom et là je je vois pas le, l'inconvénient effectivement qu'il puisse compatie compenser dans le cadre Dusan. Merci Monsieur Dantec le 192. merci monsieur le président. Je crois que nous avons eu le le débat tout le monde a bien compris. Donc c'est un amendement très simple qui vise effectivement à ce que. Les surfaces que nous mettons dans ce conte national soit réparti de façon équitable entre les régions, selon des modalités fixées par décret.

Qui le défend. Elle dit monsieur Boyer. de la consommation du foncier de l'artificialisation. En effet, la rédaction actuelle qui ne concerne que l'article 194 permet de sortir ces projets des documents régionaux, mais il reste dans le compte font dans le compte foncier national et impacteront donc de la même manière les capacités foncières du bloc local avec le poids des projets d'envergure nationale dans le fond si mobilisables. Pour la décennie 21 31 par le bloc local, qui représente 10 et et 35% de l'enveloppe restantes et une réduction de consommation du foncier entre moins 60 et moins 85% pour les élus du Bloc local avant de territorialisation. Merci donc avis de la commission sur ces neuf amendements. Permettrait de rappeler un fil rouge à partir de 2 points. D'une part qu'il est, il est toujours risqué de se lancer dans des listes. On en connaît tous les limites et surtout d'oublier certains sujets et d'autre part qu'il ne faut pas étant de manière excessive, le périmètre couvert par ses projets et rester à des projets qui par nature on ne donnait pas que dépassant le cadre d'une d'une région. Alors en ce qui concerne les amendements 62 63 de monsieur Bila qui propose de renvoyer une enveloppe nationale l'artificialisation induite par les bâtiments publics d'intérêt collectif au service public, c'est 62 ou d'exploitation agricole 63. Dire que l'enveloppe nationale doit correspondre à des projets d'une ampleur qui n'pas. C'est le cas de la région. C'est un avis défavorable. Le 41 de monsieur Longeau le 110 Monsieur avec des rédactions différentes bien sûr incluent différentes sortes d'infrastructures environnementales ou concourant à la gestion des déchets, là encore on est pas dans des projets d'dans

Nous pensons au contraire je l'ai dit précédemment, que l'État doit prendre toute sa part dans l'effort de sobriété foncière et pas seulement les régions et c'est bien le sens des modifications que la commission a apporté à l'article IV et qui sont d'ailleurs supprimés par l'article par l'amendement 205 donc c'est donc une demande de retrait sinon défavorable. Le sens de monsieur ne peut pas être adoptée, car il vise l'alinéa de l'article qui n'existe pas, sauf erreur de ma part. En outre, il demande un rapport qui est déjà prévu à l'article à la une, et à 12 du présent article et enfin de 192 Monsieur Dantec. Il me propose le gouvernement d'imputer sur les enveloppes d'artificialisation des régions celles résultant des grands projets principe auquel nous avons déjà exprimé notre désaccord c'est un avis défavorable en résumé demande de retrait sinon défavorable sur tous les amendements de la discussion commune.

Donc nous allons passer au au vote sur ces amendements. Avec un à un double avis défavorable surtout sauf. Donc un avis de sagesse sur celui de Monsieur Dantec de la part du gouvernement.

Même vote. Le 41 rectifié du président Longeau qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté le 110 rectifié de Monsieur Jeunet. La grande. le 205. Oui, alors je le retire mais j'aimerais avoir la réponse Monsieur le Ministre les gendarmerie nationale. Et retirer ensuite le sens rectifié. Une. Alors celui de Monsieur Dantec le 192 qu'un avis défavorable de la commission. Un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté. Et enfin les deux amendements identiques, le 215 rectifier bis et le 228. Double avis des frais. Monsieur Rambo retiré. Monsieur Boyer les maintenu. il est maintenu, donc je le soumets aux voix avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté À l'amendement 94 il y a personne pour le soutenir. N'est pas présenté le 211 Madame brûlant. Merci monsieur le président. Si vous m'y autorisez, je défendrai le 211 et le 212 dans la foulée. Le 211. Vise à essayer de se donner des garanties que les porteurs de projet. Intègre. Au moment même de leur projet. Les enjeux de du zéro artificialisation nette parce que depuis tout à l'heure nous évoquons. Beaucoup et c'est légitime. L'effort des collectivités. En faveur Dusan. Mais que cette dimension-là doit aussi être pris en compte par les porteurs de projets qui, comme vous l'avez dit, monsieur le Ministre peuvent être de l'appui de l'Ordre de la puissance publique mais qui peuvent aussi être des porteurs de projet privés et qui tout autant que les collectivités doivent contribuer à cet effort, donc ça c'est le 211 et le 212. Je l'ai plus ou moins évoquée tout à l'heure. Au sujet de l'amendement du gouvernement parce que autant ça été rappelé tout à l'heure par notre collègue Gremillet. Dans le texte accélération du nucléaire que grâce à cet article 4 de la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui le Sénat. Multiplie les initiatives pour que un certain nombre de grands projets d'intérêt national, voire européen n'impacte pas les régions concernées en terme de Anne mais avec une vision encore un peu restrictive au sens je j'ai cité l'exemple de l'EPR. Mais je pourrais citer d'autres exemples où pour accueillir un grand projet de ce type. Cela nécessite que les territoires développe tout un tas d'infrastructures d'accueil de transport etc. Je vais poser la question à l'envers. Que se passerait-il si un territoire, qui devaient accueillir. Une ligne ferroviaire une autoroute hein, mon père ou que sais-je. N'était pas en situation au regard de ses capacités d'artificialisation d'accueillir les salariés par exemple qui devrait contribuer au chantier. Je pense que c'est une vraie question. Et que pour l'instant elle n'a pas complètement trouver de réponse. Merci. Merci. monsieur le président. Nous avons déjà renforcé en commission là à la l'idée à 12 et la prise en compte de l'enjeu posé par l'artificialisation des sols par les grands projets qui ne peut pas être exonérés de tout effort. C'est un amendement satisfait semble-t-il sur ce point. Quant à la question de la perméabilité des sols. Elle concerne l'ensemble des projets et pas seulement les les grands projets. Et je partage sur le fond, il est vrai qu'il faudra traiter la question des services. Éco-systémiques rendu par les sols et c'est peut-être là le droit européen qu'on a évoqué tout à l'heure qui nous y amènera.

C'est un vrai sujet effectivement là aussi que que vous posez, je chers collègues le. Cet amendement là là là encore par d'une intention. En effet, que je partage mais il n'est pas possible de traiter de la même manière le projet lui-même et ses conséquences directes ou indirectes, parmi lesquels l'installation des salariés de raccordements routiers. L'idée de laisser à la région lors de la définition de ces projets. Le soin de préciser l'emprise exactes et le périmètre de ces de ces projets. Donc ce sera aussi à l'avis défavorable. Monsieur le Ministre. Avis défavorable pour la même raison que le rapporteur sur le premier et sur le deuxième pour les c'est aussi une liberté aux salariés sur l'endroit d'habiter, c'est-à-dire que si je commence à l'expliquer que j'ai un compte à part, est ce que je le fais dans la commune, qui est le siège de l'équipement. Alors que certains pour avoir peut-être envie d'habiter un peu plus loin parce que la composition du foyer, fait que l'voudra travailler la jonction d'un autre territoire, on aura une difficulté à détour et les besoins des salariés de ces projets à partir de quelle ampleur. Des projets on détermine qu'il faut prévoir les niveaux de logement et dans un contexte. Où la population française, sauf s'il y a des infos que je n'ai pas n'augmentera pas de la somme des grands projets mais se se répartira aussi en fonction de là où seront les projets d'attractivité du territoire. monsieur le ministre. Alors sur le premier déjà le sens donc double avis défavorable, y a-t-il des demandes d'explications de vote. Non donc le soumet aux voix. Qui est pour. Qui est pour. Il s'abstient. Il n'est pas adopté. 212 doubles avis défavorable, demandes d'explications de vote. Qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient. Il n'est pas adopté ensuite. L'amendement 131 rectifié.

Les grands projets, cela permet de renforcer l'éligibilité de ces infrastructures à la catégorisation de grands projets d'ampleur nationale ou européenne et d'intérêt général majeur et notamment le canal Seine Nord Europe dont les atouts en faveur de la transition écologique sont déterminants pour atteindre nos objectifs nationaux de verdissement des mobilités. Il est ainsi crucial de s'assurer qu'un tel projet d'envergure européenne ne pénalise il sera pas la région traversée pour le bien de tout le pays et de tout le continent. Merci. Avis du rapporteur sur cet amendement. donc en l'état ces retraits ou favorable. Je le ministre. Idem, étant entendu que pour le coup pour s'en Europe il y a pas de débat, on est tous d'accord. Un double avis défavorable, vous mentez. L'amendement Monsieur Domi il est maintenu, donc je le soumets aux voies. Pardon, excusez-moi monsieur Beuchere. sur le canal Seine Nord, je me suis suffisamment battue ici y compris pour les financements et c'est pas la maison têtards qui dira le contraire. Et on est je pense effectivement de manière transpartisane. À avoir été. Sur ce sujet. Monsieur le Ministre, si vous pouviez nous dire. Vraiment, clairement. Le canal Seine-Nord Europe. Sort Dusan. C'est ça qu'on attend ce soir sur ce truc-là donc, vous le dites très clairement pour que ce soit aussi clair plutôt que oui oui on a tous conscience. Monsieur le ministre. c'est que le canal Seine Nord Europe ne peut pas être imputés à la seule charge de la région des Hauts-de-France et qu'il a la caractéristique de grands projets d'envergure nationale. Si vous voulez me faire dire qui disparaît complètement. Et qu'il n'existe plus en termes d'artificialisation c'est là où on a le débat sur le compte à Paris, jusqu'où on va. Mais ça c'est un débat qui vaut pour Seine Nord Europe et pour le reste. Depuis le début il y a bien les deux lignes, qu'est ce qui est un grand projet d'envergure nationale. Le canal Seine Nord robe en fait partie. Et ce qu'il est quelque part dans les 125.000 hectares des 10 ans qui viennent ou est-ce qu'il est nulle part. En artificialisation gratuite, c'est là où on a un débat. Allez-y monsieur Arnault. réparti dans le Cantal, dans les Hautes-Alpes. Dans le Cantal et dans le Lot. Ça veut dire ça. Non mais soyons précis, et ça c'est inacceptable. Ça veut dire que ça participera à hauteur de 10 hectares par département sur les 1000 hectares dont nous parlons. Mais monsieur le sénateur. Les espèces les écosystèmes. Je veux bien plein de choses, on discute depuis le début de toutes les activités humaines. À un moment. On ne peut pas à la fois être convaincu que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Ça suppose de conserver des capacités de stockage dans les sols. Participez des inquiétudes réelles sur les difficultés de stockage liée à la sécheresse considéré que l'extinction des espèces n'est pas une fable et qu'on a besoin, collectivement, de regarder comment on les préserve et à la fin. Trouver 50 bonnes raisons de faire passer la biodiversité après ses activités d'artificialisation. monsieur Arnaud. Je suis désolé mais vous avez déjà pris la parole. Donc. Madame Cukierman.

je crois qu'il faut avoir la responsabilité effectivement des évolutions. Climatiques et environnementales sans non plus alimenter un scénario catastrophique qui viserait à ce que nous fassions plus rien parce que y compris, on le sait. Et et l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité. C'est aussi cette force. Non pas à nier ou à mettre la poussière sous le sous le tapis mais a aussi à certains moments donnés par. Par l'Intelligence humaine donc par la recherche par. L'industrie par la production. Des débouchés scientifique de trouver des réponses et des capacités qui vise à la fois à permettre la la présence humaine et à préserver la planète même si effectivement là encore à l'échelle de l'humanité. Cela n'a pas toujours été le cas et donc la question n'est pas de de nier ce qui a pu fonctionner ou pas. Mais vous voyez. Je crois que on arrive là aussi avec un une vraie difficulté, c'est qu'on fait, ben voilà ce qui est en train de se passer c'est que à la fin on réouvre des guerres territoriales. On a, on enlève le vrai débat de stratégies nationales de souveraineté. Dans tous Dans tous les sens du terme. Et où on va effectivement renvoyer et ce que quoi, un discours de chiffonniers. Parce que bientôt on va acheter à la grattage et puis chacun prendra le projet qui veut pour mieux se le répartir et ben aménager un pays, je pense que ce n'est pas ça. Aménager un territoire, cela n'est pas ça. Et on peut très bien aujourd'hui avoir une vision qui vise à protéger les espèces et qui permet tout de même la la l'installation de grandes de grandes infrastructures sans qu'il y a des territoires qui soient perdant-perdant. Bonjour. Oui, monsieur le président. Je je j'ai sursauté à la réponse du ministre. Aux interpellations de messieurs Bachere et Arnaud quand vous avez justifié Monsieur le Ministre, le fait de redistribuer globalement l'enveloppe entre guillemets car que le canal Nord prendrait parce que vous avez justifié cela par la nécessité de préserver la biodiversité. Le but, l'un des deux buts peut être le but 1er du canal Seine-Nord c'était pas déjà quand même un but écologique. Bon alors honnêtement je. Vous êtes dans une double contradiction enfin je je comprends vraiment pas, honnêtement je comprends pas votre raisonnement, je le comprends pas. Bien chers collègues nous allons Monsieur Salmon. Merci monsieur le président. C'est le ministre, mes chers collègues. Je crois qu'on, on en revient. À notre notion des urgences qui n'est pas partagé ici. Clairement, on est devant des défis incroyables hein j'entends bien ma collègue Cukierman qui dit que ben on peut penser que la technologie que la science. Va être suffisante. Pour affronter les défis de demain et que ça nous évite peut-être de nous pencher trop sur la nécessité d'efficacité de sobriété de société. Je pense clairement que nous ne sommes dans de telles urgence qu'il faut agir sans tarder et que c'est une question également de de solidarité d'avenir commun. Nous avons. Une biosphère. Nous avons une planète nous n'en avons pas de rechange et clairement continuer à mettre le paradigme de l'économie. Au-dessus de notre environnement. Je pense que c'est une erreur, une erreur colossale, et on le voit bien les année après année. L'homme ne peut s'affranchir de son. Environnement et de la planète et donc il y a un moment, soit on pose les choses. Et on essaye d'avancer ensemble, sans essayer effectivement de se battre comme des chiffonniers, avec des petits entre guillemets et des petits échos d'égoïsmes territoriaux. Je pense qu'il faut aller il faut aller de l'avant, clairement Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire que à un moment soit en avance. Soit on continue comme avant. Oui, merci Monsieur le Président. Lorsqu'on parle de protection de la biodiversité. Il y a aujourd'hui sur le territoire national. 58 parcs naturels régionaux. Et on. Nationaux. Qui représente une superficie en terme de de d'hectares. Relativement importante et dont l'objet principal de ces parcs aussi bien naturels régionaux que que nationaux et la protection de la biodiversité. Et les moyens financiers qui sont mis pour la protection de cette biodiversité, que ce soit des moyens des conseils régionaux, des conseils départementaux, ce sont des donc les Les impôts des contribuables français qui, qui participent de manière. Importante à la protection de cette biodiversité, parce que c'est le un des objectifs premiers. Un des objectifs fondamentaux. La protection des biens de la biodiversité de ces différents parcs. Donc. Effectivement, lorsqu'on a des projets d'envergure nationale. Qui ont. Un impact économique un impact d'emploi parce qu'il faudra bien qu'un moment donné on parle quand même un petit peu de la vie de nos concitoyens, qu'on parle de l'emploi que l'on parle de l'économie de notre territoire et qu'il s'agira, je pense, de trouver un juste équilibre. Parce que je pense que le effectivement le coeur, je vous le disais tout à l'heure de la proposition qui est faite aujourd'hui, c'est de trouver un juste équilibre, qu'il peut y avoir entre l'impact. Les objectifs environnementaux qu'il faut qu'on recherche certes, mais aussi l'activité économique de nos territoires et la vie nos concitoyens et on ne pourra pas rester toujours sourd à ces objectifs là qui me paraissent importants. Chers collègues, je demande à nos collègues écologistes. De bien prendre la mesure qu'on est tout ce qu'on sait en tout cas pour notre groupe. De la gravité de la situation en terme de réchauffement climatique et biodiversité. Mais chaque fois qu'on réindustrialiser la France. Pour éviter qu'on externalise en Chine ou dans d'autres pays. Des produits qui vont être plus polluant et qui vont avoir des conséquences dans les transports. On contribue à l'équilibre global de la planète et à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc nous avons besoin. Évidemment on ne va pas re-localiser pour polluer comme des malades en utilisant les technologies d'aujourd'hui, elle est savoir-faire d'aujourd'hui et même en anticipant. Donc on ne peut pas considérer que prendre en compte la, la pression, j'ai bien entendu ce que dit le gouvernement, qui tend à dire tout ça va rentrer dans le, dans le cadre je l'espère. Mais je souhaiterais qu'on soit plus précis sur la vérité des prix si je puis dire en termes de mettre de, de d'hectares consommer pour cette réindustrialisation. Et puis deuxièmement. Moi je pense qu'il faut être efficace. Et pour le coup pragmatique. On peut toujours décider qu'il a des dispositifs qui vont naturellement parce qu'on les aura voté s'appliquer. Et croire que la contrainte la sanction machin. Puis quelques années après on se rend compte que ça passe pas. Parce que l'opinion ne veut pas parce que les, les élus refusent parce que les réalités s'imposent. Et j'observe. Que par exemple, le gouvernement allemand.

Et j'entends pas. Les écologistes allemands hurler au scandale. Donc personnellement je dis il va falloir qu'on trouve l'équilibre. Et cette année il. Le il faut conclure et en particulier sur cette histoire de Zan que je crois quand même assez mal parti mais tentons de le réussir. Merci monsieur Sautarel. OK pour faire remonter mais pour faire redescendre je je ne vois pas comment on peut faire redescendre, parce que les les inégalités. Aujourd'hui, elles sont multiples. Il si on veut rechercher soit des possibilités de renaturation ou de développement sur les friches que vous évoquiez tout à l'heure sans doute que les friches ne sont pas non plus réparti de manière équitable sur le territoire et donc ça peut être un critère. Par rapport à ce compte. National qui pourrait être utilisé en tout cas je autant l'objectif du nationale il est indépassable, autant il ne peut pas redescendre sur les territoires comme ça semble être imaginées. Et ce n'est pas de de l'égoïsme sur nos territoires vous il y a des territoires ruraux. Pour l'instant j'ai j'ai j'ai parlé quand je suis intervenu de manière assez globale mais en tant que sénateur du Cantal. mon principal souci d'artificialisation des sols. C'est les blocs béton si on veut nous poser des éoliennes et ça nous réjouit pas vous savez hein donc je, je pense que de ce point de vue là, on ne cherche pas à avoir des surfaces artificielles artificialiser supplémentaires et je voulais juste à cette heure un peu tardive mais il me vient une image parce qu'on voit bien qu'on est sur des sujets de complexité par rapport à ses objectifs de développement durable, l'environnement et, et donc par rapport aux contraintes multiples et et parfois paradoxal que l'on peut rencontrer comme Madame Lienemann vient de le rappeler. On peut prendre cette image d'un bocal. Si vous mettez des galets dans un bocal et qu'on vous pose la question, vous dites il est plein. Mais vous pouvez continuer à mais du sable dans ce bocal et vous dites il est plein et après vous pouvez mettre de l'eau et il est toujours en et et il est toujours plein et ça déborde pas donc il faut qu'on arrive à cumuler nos trois objectifs sans doute de développement durable, de la même manière. Merci.

Merci, monsieur le Président, j'ai failli rester sans voix. Après la brillante démonstration de notre collègue Sautarel sur son bocal ces galets le sable et l'eau. Néanmoins je reprends mes esprits pour présenter cet amendement. Qui se rapproche de ce que vous disiez monsieur le ministre et j'étais assez d'accord avec vous sur les difficultés qu'on observe des aujourd'hui dans un certain nombre de territoires pour obtenir des permis de construire et mener à bien un certain nombre de projets et comme je vous parlais des des débats auxquels j'assiste sur le terrain pour la préparation d'un pays lui je suis marqué par les réflexions qu'on commence à entendre sur, en particulier l'accueil de d'activité logistique sur les territoires. Les élus locaux disant bah puisqu'on nous impose Lausanne. Il faut maintenant qu'on choisisse le type d'activité qu'on veut accueillir et et pourquoi accueillir des activités qui consommerait beaucoup de foncier, alors qu'on pourrait privilégier d'autres activités qui accueillerait peut-être plus d'emplois Ses activités logistiques sont tout de même très importante pour notre économie et c'est pourquoi. Je mets au débat cet amendement pour. Insérer à l'alinéa 8 après le mot industrielles. Les mots et logistique. Pour pouvoir intégrer donc ses ses activités dans l'enveloppe nationale. Ce ça pourrait être de types de zones logistiques à la fois les unités logistiques qui sont directement rattachés qui valorise les infrastructures d'ampleur nationale cité au ah et oh c'est de l'article IV ses implantations logistiques rattaché à ces projets sont en effet indispensables à leur bon fonctionnement et à leur utilité concrète et puis deuxièmement, les unités logistiques qui, au même titre que les usines et souvent en complément, voire au service des usines concours à la transition énergétique ou à l'indépendance nationale comme les zones logistiques, liés à la réindustrialisation, celle des chantiers des nouvelles centrales nucléaires ou les stations d'avitaillement d'énergie alternative au diésel fossile. Monsieur le président. Et chers collègues qui va finir par penser que je lui en veux donc avec mes avis défavorables mais ce n'est pas du tout le cas. Fabien. Néanmoins, alors c'est comme pour les listes les critères plusieurs des critères plus il y a de risques de d'oubli et. Et tous les risques afférents à trop de précision et par ailleurs. Pour pour moi c'est vraiment la fonction du sera d'être. D'appréhender les sujets de logistique et d'unité de logistique et donc d'appréhender précisément l'emprise de ces de ces projets leur surface

qui est pour. Contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté cet amendement identique en discussion commune le 40 rectifier Monsieur

Il conviendrait que la liste des projets concernent ne soit pas trop restrictive et qu'elle puisse notamment inclure des projets d'activité économique d'ampleur nationale, voire européenne. Et ce, conformément aux objectifs affichés de ré-industrialisation de notre pays dans des secteurs stratégiques, je pense notamment à Airbus à Toulouse, c'est le projet qui est présenté ici. Allô. Merci monsieur sûrement le suivant. Pour défendre l'excellent amendement de monsieur Cadec mais qui a été excellemment défendu par Monsieur Bonhomme. Si Madame Micouleau le 70 districts. Merci monsieur le président. Moi je voudrais quand même insister sur le fait que sur les 32 métropoles françaises. N'ont contribué depuis 2009. Ils n'ont utilisé que 1% d'artifice d'artificialisation. Du pays et reprendre l'exemple d'Airbus en tant que Toulousaine. S'il est mis trop de bâtons dans les roues de l'entreprise elle-délocalisera et la délocalisation veut dire moins d'emplois et surtout pas de création d'emplois. Merci.

Communs en tout cas qui vise finalement. À s'assurer de pas de ne pas renvoyer la responsabilité uniquement au niveau des collectivités mais mais bel et bien d'inclure les projets répondant à des enjeux de souveraineté. Nationale et européenne dans une enveloppe nationale. Je crois que ça a été dit à travers divers exemples on pourra en citer énormément, il y a bien évidemment derrière des enjeux. Industriels, il y a des enjeux de richesse de production il y a des, des enjeux d'emplois. Il a des enjeux d'aménagement du territoire. S'il y a des femmes et des hommes qui vivent sur un territoire il y a deux il y a donc des enjeux pour les nourrir, il y a donc une enjeu à avoir des territoires aménagé sur lequel il y a une agriculture qui soit vivant et qu'qui soit nourricière. Bref, il y a tout un écosystème positif. Oui positif et vertueux à préserver et en tout cas elle est le sens de notre amendement. Merci monsieur le président, qui est identique. À celui de ma collègue qui l'a excellemment défendu, je voudrais juste ajouter. Que en la matière, il ne faudrait pas tomber dans le pli très français qui est d'avoir des bonnes intentions. De se mettre beaucoup de carcan et au final, finalement de repousser un peu plus loin, la poussière et en la matière d'aller produire à l'étranger parce que finalement qu'est-ce qu'on y gagnerait. C'est ce que Madame Lienemann disait très très bien tout à l'heure si effectivement on a les meilleures intentions du monde et que on empêche toute activité en France et que cela conduit à les produire à l'étranger de réimporter ensuite sur notre territoire, on n'aura rien gagné ni pour l'emploi en France, ni pour nos concitoyens ni pour la planète. Monsieur. Le suivant défendu monsieur le président. Défendu et monsieur Corbizet dernier défendu. Donc sur ces 7 amendements identiques. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président. Monsieur le Président. Tous ces précisions paraissent fort utile et ce sera un avis favorable. Je suis heureux que Monsieur soit auteur d'un amendement. Favorable de la commission, monsieur le ministre. Comme je l'ai évoqué cette liste. Elle fera l'objet d'un article spécifique dans le cadre du projet de loi industrie verte, je me remets à la sagesse de l'Assemblée, parce qu'on partage la philosophie qu'il faut intégrer sur le. À partir du Triel mais la formulation. Elle est trop vague. À ce stade pour pouvoir justifier demain. Du fait de savoir si les projets relève de cette souveraineté nationale ou européenne ont soit ça commence et ça s'arrête où tout ce qui est pas alimentaire peut pas par exemple être considérées comme faisant partie de la souveraineté tout court. Ou alors ça veut dire que le Champ de ce qu'on élargie et de ce qu'on sort devient tellement grand qu'on se retrouvera avec une difficulté sur les trajectoires de compter à part. D'où le fait que je pense qu'on a besoin de ce travail un peu plus précis des commissions sous forme d'amendement d'appel avant les échanges. Je pense que ça permet au moins de rappeler que la dimension économique doit être intégrée. Dans les assouplissements aux trajectoires. Bien, vous avez entendu les deux avis. Donc je vais soumettre ces cet amendement identique. Oh on voit qui est pour. Qui s'abstient.

Et si vous passez de droite à gauche, je ne peux pas vous retrouver. il a il a il a dit défendu pour celui-là il est défendu monsieur Bachar dit défendu. Alors allez-y, allez-y, allez-y. Ah ben quand même. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En France 2 tiers des 36.000 communes sont exposées à au moins un risque naturel glissements de terrain inondations avalanches et on sait que le dérèglement climatique amplifiera ces phénomènes. Et le nombre de territoires concernés. Le code général des collectivités territoriales mais à la charge du maire titulaire des pouvoirs de police municipale, une obligation de prévention des accidents mortels de toute nature à travers la réalisation de paravalanches de dit ou encore de murs de soutènement. En l'absence d'indication contraire dans la loi climat et résilience les travaux nécessaires constituent des opérations artificialiser les sols qui seront décomptées des droits à construire des communes malgré leur intérêt général évident et leur caractère absolument indispensable aussi. Cet amendement a pour but d'intégrer de la liste des projets de construction d'aménagement d'infrastructures présentant un intérêt général majeure non comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation tous les travaux en lien avec la protection des populations contre les risques majeurs et naturel. Je vous remercie. monsieur le président. Chers collègues, la commission. Bien évidemment. Consciente de l'importance parfois vital. Du sujet évoqué mais au niveau local et donc n'entrant pas. Pour nous dans la catégorie des grands projets autres. C'est un retrait sinon défavorable. Monsieur le Ministre. Même avis donc un double avis défavorable, je le soumets aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 191 Monsieur Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'objectif de cet amendement et de restreindre les critères permettant de considérer comme projet, projet d'ampleur nationale européenne. Les projets internes régionaux. Il est proposé donc de supprimer ce terme en effet aucune estimation n'a été faite de cette catégorie. Une telle disposition risque d'inciter les régions à inclure dans le Comte spécifique nationale des projets qui ne sont pas de cette ampleur. Les projets interrégionaux doivent être pris au compte en compte au niveau des régions concernées au prorata des espaces consommés par chaque région et comme il me reste un petit peu de quelques secondes, j'en profite pour répondre à la petite attaque perfide contre contre l'éolien très rapidement. Les blocs d'éoliennes. Effectivement s'il y a du béton, mais il faut savoir que ça représente 0,5% du béton coulé chaque année en France qui est con, c'est qu'il est pour l'éolien et que le projet Cigéo. Je sais bien que vous adorez quand même le nucléaire. 6 millions de mètres cubes. Cela représente l'équivalent de 10.000 éoliennes, c'est simplement pour vous donner un petit ordre de grandeur. Il faut savoir de quoi on parle. Monsieur le rapporteur. Sur cet amendement. Monsieur le président. C'est un amendement qui supprime la possibilité de qualifier des projets d'infrastructures inter-régionales en tant que grand projet. Pourtant l'inclusion de ces projets souhaitable afin d'et d'éviter une interprétation trop restrictive de la notion. D'infrastructures nationale une ligne à grande vitesse traversant deux ou trois régions peut en effet paraître être de très grande ampleur, justifiant son décompte en dehors des comptes fonciers régionaux sans pour autant être une infrastructure nationale sera un retrait sinon des Favorable. Le ministre. Même avis donc un double avis défavorable sur cet amendement Monsieur Dantec. Oui, sans être trop long. J'ai j'ai bien entendu les arguments sur les sujets précédents mais la. mais la. Ça veut dire qu'à la limite une route départementale qui passerait entre 2 régions c'est de l'intérêt régional un pont. C'est de l'intérieur on peut mettre énormément de choses et là on sort vraiment vraiment du débat précédant. Là c'est vraiment. On s'organise pour essayer de passer le maximum de choses sur le camp national et faire le minimum d'efforts sur les territoires. Donc je trouve que vraiment. Là on joue un jeu extrêmement dangereux et compris on décrédibilise le débat sur les vrais enjeux de ce qui doit être mis dans le Comte nationale parce que la, la liste va être sans fin de tout ce qui passe d'une région à l'autre. Bien donc je soumets l'amendement. O voir. Qui est favorable à cet amendement. Qui est défavorable. Il n'est pas adopté le 28 rectifié monsieur Arnaud. Oui, monsieur le président, il s'agit simplement. De rajouter un mot, un petit mot. Le mot international pour intégrer dans l'enveloppe nationale les grands projets d'envergure nationale, comme c'est indiqué dans le texte ou européenne, mais il y a également des projets ah coopération multiples et pas simplement dans le cadre européen, je pense aux projets en cours de réalisation militaires dans les Bouches-du-Rhône, également dans les Alpes Provence ou encore les installations astronomiques et inter-Chéreau métrique du plateau de Bure dans les Hautes-Alpes, donc je pense que dans d'autres territoires de France on a des projets en coopérations multiples qu'il s'agit effectivement puisqu'ils sont d'intérêt supranationale et même supra-européen d'intégrer dans l'enveloppe nationale par ailleurs j'en profite puisque j'ai la parole pour demander à monsieur le Ministre, s'il avait la gentillesse éventuellement de nous éclairer sur un point qui me fait défaut. C'est de savoir de quelle manière les voisins. Belges. Allemands, italiens. Espagnols appréhende la question Dusan à leur échelle, parce qu'on est également dans une économie européenne et il nous semble important de savoir de quelle manière se localise les activités qui, comme vous le savez, peuvent venir en France et on en est heureux parce que ça crée à la fois de développement économique, ça crée de l'emploi, ça crée une dynamique également parfois de transition sur un certain nombre de modalités de production de nouvelles énergies. J'espère que ce que nous sommes en train de faire 2 retricoter peut être à la maille du du Sénat ne sera pas un handicap complémentaires sur la compétitivité nationale et sur la souveraineté nationale. Merci de votre réponse. Merci. Avis de la commission sur cet amendement. Le le président c'est une proposition intéressante importante et raisonnables. Ce sera favorable. Monsieur le Ministre. Je vais pas faire un, un temps de droit comparé. Pour le sénateur Arnaud seulement pour dire que la date de 2050 dans tous ces pays elle vaut comme trajectoire de zéro artificialisation nette avec ensuite des différences qui s'explique aussi par les compositions territoriale mais la plupart du temps en tout cas pour l'Allemagne c'est bien les Länder qui se retrouve à être l'échelon pivot qui fait en sorte ensuite. Que le dispositif parce La proposition qui est faite par le sénateur Arnaud comme beaucoup d'autres. Elle participe à ajouter et assure ajouter des catégories et à la fin. Ça rend d'autant plus compliqué le discours que nous avons sur le comté à part et ça rendra d'autant plus complexe le fait d'arriver à trouver des équilibres entre les 2 assemblées. Donc pour cette raison, je ne suis pas favoris. Bien donc sur cet amendement 28 rectifié bis, un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient.

Sur le 132 ce le président. Le 132 oui. Oui tout à fait. Merci. Alors en fait sur ce sujet. On nous en serions Émile l'avis du gouvernement. L'avis du gouvernement est défavorable. Et donc l'avis de la commission. il ne paraissait que la la la question posée était était importante. Concernant précisément les les projets faisant l'objet d'une décision d'exécution donc ce, ce qu'on peut en savoir plus sur le défaveur caractère défavorable. De l'avis du gouvernement Le gouvernement avait synthétisé dans l'amendement 181 qui a été repoussée par cette assemblée, la procédure sur laquelle elle s'appuyer, qui prévoyait une liste qui prévoyait un arrêté ministériel qui prévoyait un dispositif de concertation avec les collectivités territoriales pour la partie publique et qui prévoyait un dispositif remis dans le l'industrie verte, je peux déposer un sous-amendement qui consisterait à faire revenir l'amendement 180 sous une autre forme pour qu'on abrège le débat sur la totalité de l'article IV mais quelque chose me dit que j'aurais un avis défavorable du rapporteur dont je ne propose pas. Mais nous restons dans notre cohérence. Bien, donc nous allons soumettre aux voix cet amendement. Qui est pour. Sagesse. Qui est contre. N'est pas adopté. 3 amendements. Et un sous-amendement qui font maintenant l'objet d'une discussion commune. D'abord 3 amendements identiques, le 52 rectifié Monsieur Étienne Blanc. Oui. Monsieur le président. Et je je me demande si cet amendement. Et ne tombe pas avec l'adoption du 180 rectifié. Non. Et. Je sais pas. Monsieur le rapporteur. Est ce que. Je le présente le 180 je je le présente telle alors. Oui, allez-y, allez-y, présentez le. Oui. Il s'agit. De de d'aborder la question des des grands ports maritimes. Et de considérer. Qu'il faut pas seulement prendre en considération le port maritime lui-même mais la circonscription administrative du port maritime. Telle qu'elle est précédents dans le code des transports qui précise qu'un grand port maritime peut intervenir directement sur l'étendue de sa circonscription administrative au delà du domaine portuaire au regard des des interactions générée par ses activités. C'est tout l'objet de cet amendement. Merci le 170 rectifié madame Canayer. Oui, merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, 3 arguments en faveur de cet amendement identique à celui de mon collègue blanc le 1er c'est que nous sommes dans le cadre d'une limitation géographique, celle de la circonscription portuaire effectivement d'inscrire les opérations d'aménagement réalisé au sein des grands ports dans. Le compte foncier national. C'est un enjeu qui dépasse l'enjeu strictement local parce que pour les grands ports maritimes comme évidemment ceux de l'axe Seine. Aropa Le Havre, Rouen et Paris c'est un enjeu de souveraineté économique et industrielle française puisque c'est pour permettre le développement Fax face à la concurrence des grands ports européens, notamment ceux d'Anvers et c'est aussi 3ème argument un enjeu. de stratégie et de développement environnemental puisque c'est permettre tous les projets de décarbonation de l'économie, tous les projets industriels qui vont dans ce sens. Donc c'est tout l'intérêt de cet amendement. Merci enfin le. Monsieur Mandelli.

merci Monsieur le Président. Cet amendement qui est identique a d'ores et déjà été défendu mais je voudrais simplement rappeler avant le sous-amendement puisque qui répare un oubli puisque j'ai oublié d'intégrer les les ports fluviaux proprement dit dans le dans l'amendement. Simplement se rappeler qu'au,

Que ce qui a façonné à la fois nos paysages et notre pays globalement en terme de développement et de sa richesse, sa création de richesse, ce sont nos rivières nos fleuves et nos façades maritimes toutes les métropoles que nous connaissons se sont développées sur ces axes majeurs qui étaient. Les fleuves et et qui plus est ensuite avec les les ports dans et leurs estuaire et il faut se le rappeler parce que à une époque. Ici comme ailleurs il n'y avait pas ni camion. Ni avions. Ni ferroviaire pour acheminer les les les hommes et les marchandises et ça se faisait évidemment travers des ports. Et et et des fleuves et que, au moment où. L'économie. Est de plus en plus mondialisées. De plus en plus de transport maritime, plus de 90% des marchandises transportées par la mer, hé bien il est important que nous puissions préserver cette capacité ses poumons et moins économique pour notre pays si on veut développer le transport fluvial le doublé, c'est l'objectif. Eh bien je je pense que nous devons adopter ces amendements nos rivières et nos fleuves ont donné les noms de nos communes de beaucoup de nos départements. J'ai pas tous les citer. Et beaucoup de, de nos régions donc il il faut à l'oublier c'est. C'est l'essence même du développement de notre pays. Et donc Madame Loisier pour le le sous-amendement que vient d'évoquer rapidement monsieur Mandelli. Madame, monsieur le président, monsieur le ministre, il s'agit juste donc de préciser la la référence juridique on y incluant les les ports fluviaux merci. OK. Merci monsieur le rapporteur. Sur ces. Trois amendements sous sous-amendé, avec les ports fluviaux. Oui, monsieur le président. Alors ces trois amendements traite de la question des circonscriptions administratives des grands ports. Alors l'amendement 170 Canayer complètent la liste des critères. En dissipant un doute qui s'était fait jour les projets d'ampleur nationale ou européenne doit pouvoir devrait pouvoir inclure des projets me menés non pas strictement dans le périmètre des grands ports même mais aussi au sein des circonscriptions administratives.

pas pu être examiné par la commission. Spéciale. Je ne me donnerai donc un avis personnel mais regrettant qu'on n'ait pas pu en discuter vraiment et de fait. Faut-il voir dans le fluvial du National ça aurait mérité. Une vraie des discussions là. En tout cas l'amendement de 182 monsieur Mandelli comme si le 170 inclus. Parmi les critères des projets d'ampleur nationale européenne. Les ports mentionné au code, c'est-à-dire les grands ports maritimes et fluviaux maritimes relevant de le, Et je rappelle que nous parlons des projets d'ampleur nationale européenne qui aura un impact tellement vaste qu'il est naturel de décompter leur artificialisation au plan national ou régional. Je sais donc il y a beaucoup de regrets que je demanderai le retrait de ce sous-amendement 262

Nous sommes défavorables à ces trois amendements pour une subtilité qui est la notion de circonscriptions. Dans l'amendement du gouvernement. Tous les projets des grands ports. Porté par les grands ports faisait l'objet. D'un comté à part mais les projets qui sont à l'intérieur de la circonscription, ils peuvent ne pas être porté par les grands ports. Et donc on peut avoir des projets qui ne participent pas directement l'activité industrielle comme par exemple l'activité. L'installation d'un restaurant d'un restaurant à l'intérieur de la circonscription du grand port si on prend la notion de circonscriptions elle rentrerait donc comptés à part, c'est pour ça qu'on préférait la porte d'entrée qui soit celle du projet des grands ports maritimes ou fluviaux et que c'est ce qui explique la rédaction qui était dans l'article 180 du gouvernement plutôt que la référence à la circonscription. Qui peut doubler ou tripler la surface des hectares qui sont concernés et nous on considère que ça doit pas être le territoire mais bien. L'impulsion en l'espèce du grand port qui doit caractériser le caractère d'envergure nationale. Donc un avis défavorable du gouvernement est favorable mais avant qu'on passe au vote peut être Madame loisirs, vous devez nous dire si vous maintenez le sous-amendement compte tenu la remarque du rapporteur. Si monsieur le rapporteur. Ma porte là l'assurance qu'effectivement les ports fluviaux sont bien intégrés les porcs sur le Rhin, Strasbourg, Mulhouse, j'y vois aucun inconvénient mais ce serait sinon juste dommage de ne pas les intégrer vu. Les l'enjeu stratégique sur les ports fluviaux. On me confirme donc je le retire. Non non mais il faut, il faut tirer. Je ne suis pas en mesure de le confirmer. J'ai juste relever des grands ports maritimes fluviaux maritimes relevant de l'État, c'est tout ce que je préfère à ce stade, dont je regrette fortement qu'on aurait ben voilà pas pouvoir en dire plus, qu'on n'ait pas pu discuter. En commission. Bien. De toute façon donc là le sous-amendement est retiré. Donc je vais soumettre aux voix en même temps les trois ces trois amendements avec un avis défavorable du gouvernement est favorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils sont adoptés, excusez-moi. Nous passons 224 rectifié monsieur Delcros. Alors mon amendement ne modifie pas l'article IV. Telle qu'il a été amendé au cours de de la discussion qui viennent de se dérouler. Simplement il apporte une précision

Et Monsieur le Ministre, nous a indiqué tout à l'heure que la dimension économique était évidemment à prendre en compte et je considère que l'activité agricole et agroalimentaire relève bien de la dimension économique. Monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le président. On est tous évidemment favorable à la souveraineté alimentaire. Mais en l'état. Dans le cas Dusan c'est une notion qui me paraît difficile à à délimiter. Il y a des il y a à définir qui relèvent plutôt de l'organisation générale secteur agricole et agroalimentaire plutôt que précisément dans un débat de 2 De retrait sinon défavorable. Monsieur le Ministre. Donc. Idem, donc double avis défavorable. Demande de retrait, vous mentez. L'amendement. Oui je je le retire simplement cela me permet de marquer le fait que dans des réflexions qui seront conduits à l'avenir on n'oublie pas tout le volet agricole c'est aussi une question d'équilibre de traitement des territoires et des départements. Merci monsieur le laïc est retiré donc monsieur Blanc le 151 rectifié. Oui, merci Monsieur le Président. L'article 3 du texte. Et énumère différents types de projets qui sont appelés à être qualifié d'ampleur nationale ou européenne. Mais cet article 3 n'évoque pas les abords des ont prise. Et on peut penser que certains équipements ou aménagements qui sont connexes à l'infrastructure concernés sont indispensables de l'emprise. Et qu'il n'apporte pas au territoire intéresser davantage de plus values Didier que le projet d'infrastructure lui-même c'est l'exemple. Du poste de transformation électrique d'un parc éolien en mer ou d'une centrale. Nucléaire et ce qui illustre parfaitement cette idée, donc ces équipements ou aménagements connexes représentent une emprise foncière significative et si cette emprise est comptabilisé dans la consommation dans la consommation d'espace du territoire. Ils peuvent grever totalement ses capacités de développement. C'est tout le sens de cet amendement. Monsieur le rapporteur. Amendement. Dont le sujet est important mais qui me paraît relever des des sera tête donc ce sera retrait sinon défavorable.

Merci monsieur le président, alors. Cet amendement concerne ce qu'on peut appeler les artificialisation externe c'est-à-dire les parts d'artificialisation qui sont délocalisées délocalisées entre guillemets. Par certaines régions vers d'autres territoires. Je m'explique, dans mon département de l'Oise. Nous accueillons entre guillemets des déchets inertes, qui viennent de chantier du Grand Paris. Grand Paris. Ça fait une double peine parce que. C'est pas forcément bien accepté par les populations locales et si en plus ça aboutit à amputer la part. 0 artifice socialisation nette du territoire d'accueil il y a une véritable injustice. Alors concrètement le. Présent amendement il vise à prévoir que les artificialisation résultant de projets destinés prioritairement à satisfaire les besoins d'une région. l'Île-de-France. Autre que celle où sont implantés les Hauts-de-France puisse être au moins en partie imputé. À la région entre Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, alors à mon collègue Olivier Paccaud. C'est, c'est un sujet que. Dont on a parlé. Que je comprends absolument. Mais. Ce qui, ce qui nous interroge c'est c'est la chose suivante, c'est que cette mutualisation inter-régionale précisément qui qui leur donnerait à ce que, c'est ce que c'est l'État, est-ce que c'est l'État qui leur donnerait précisément aux régions que concernés d'inscrire les projets dans leur sera tête. Qui était le cas, c'est une injonction qui paraît difficile à accepter, à faire accepter par par par les régions. Donc l'intention. Je la comprends parfaitement mais qui ordonne. La discussion interrégionales.

Je suis sur une position qui est proche de celle du rapporteur mais qui va un peu plus loin, pourquoi s'arrêter à ce moment-là aux contraintes interrégional à l'intérieur d'une même région. Un département qui accueille un équipement d'intérêt régional et qui se retrouve à devoir limiter sa propre capacité. D'artificialisation parce qu'elle rend un service La seule intercommunalité qui accueille un site d'intérêt départemental pour le compte de tout le territoire. Donc on voit bien qu'à la fin on aura toujours une difficulté si on. Descend trop bas cet article IV. Il est théoriquement sur les grands projets d'envergure nationale. Il faut qu'on accepte qu'il y ait une part de solidarité de partage comme on a envie d'ailleurs tous, quelles que soient les échelles

Et pourtant le Grand Paris n'a pas la place en Île-de-France pour accueillir ces déchets. Et donc, forcément, faut aller chez le voisin. Et ça c'est pas tout à fait acceptable. Vous pouvez le comprendre. Donc pour nous, et il y en a effectivement dans le canton d'Olivier Paccaud comme dans le bien et plus largement dans l'Oise. On est à des endroits comme il y avait des grandes carrières dont on fait de belles pierres qui font la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bien dans ces carrières, on va artificialiser au-delà, notamment pour mettre les déchets du Grand Paris et j'ai encore correspondu avec les grandes entreprises de bâtiment et travaux publics et. Je les citerai pas, mais enfin il y a il y a tout, il y a 3 grands groupes, donc ça va on peut. On les a tous vus, ils sont effectivement tous en train de nous dire on met nos déchets inertes dans l'Oise. Et ça couvre des surfaces. Importantes. Très importantes. c'est un vrai sujet. Moi je pense que ça vaudrait le coup de voter le texte pour qu'il soit revu en CMP, voire un peu avant ce qu'on en fait mais c'est quand même bizarre que on nous a refusé le Grand Paris. Dans l'Oise. On peut avoir à avoir toutes les mauvaises conséquences. allons nous allons Monsieur le Ministre. Je sens la tentation de réécrire la loi notre la loi MAPTAM de revenir sur les territoires. je pense que c'est la bonne heure pour le faire et et que c'est le moment d'en profiter pour se mettent d'accord sur un certain nombre de sujets qui ont été mal calibré sur le plan national ou régional. passer, oui nous allons passer au vote sur cet article. Monsieur, monsieur, monsieur le président. Excusez-moi, je maintiens mon mon article. Simplement, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de solidarité c'est c'est le mot que vous avez utilisé, il ne faut pas qu'elle aille toujours dans le même sens, parce que là dans, dans le cas précis des déchets du Grand Paris et la solidarité, elle va que dans un sens donc franchement qu'il y ait une alors peut-être que mon amendement n'était pas assez précis quand effectivement à l'autorité émettrice. Du ou à la décision mais objectivement il y a quand même une vraie question qui se pose, il y a une vraie question de de justice et et il y a pas que l'Oise qui est concerné. Il y a pas que le Grand Paris. sont. Que pour limiter les émissions. La maire de Paris est temporairement décidé de garder une partie des déchets à l'intérieur de la capitale plutôt que de faire en sorte de les envoyer vers l'Oise. Nous, nous allons passer au vote sur cet amendement. Donc avec un avis défavorable du ministre et un avis. Défavorable. Pas loin de la sagesse. Je sais pas trop ce que ça veut dire mais. C'est le président, je m'en tenir à la commission il faut être sérieux, c'est une commission spéciale, elle a émis un avis donc je vais m'arranger d'ailleurs cet avis après j'ai dit tendance sagesse parce qu'on a besoin d'être éclairé. Il y a des sujets qu'il faut travailler, ils vont certainement revenir donc je maintiens l'avis initial initial qui est plutôt défavorable, donc nous passons au au vote sur cet amendement 243 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Le 154 rectifié monsieur saumon. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, le présent amendement entend prendre en compte la situation spécifique des projets d'énergies renouvelables de faciliter l'application des principes de j'sur économe de l'espace mais aussi le développement des ENR dans le cadre de pour répondre à la souveraineté énergétique dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique. La la guerre et les conséquences de la guerre en Ukraine, avec les conséquences géopolitiques que nous connaissons et notamment les circuits d'approvisionnement des produits énergétiques fossiles produits pétroliers. Le gaz naturel et l'augmentation de l'énergie électrique cet amendement vise à accélérer la production des ENR éolien ou le photovoltaïque ou encore méthanisation selon les potentialités territoriale sans amputer celle foncières nécessaires au développement d'infrastructures de logement ou d'activités industrielles de chacune d'entre elles. Si ça n'est pas le cas. Monsieur le ministre, est-ce que l'État va s'appliquer les mêmes règles qu'il impose aux collectivités, là où la consommation n'a-t-elle pas été économe de depuis 10 ans je pense particulièrement au département de la Somme, où nous avons 742 éoliennes qui sont installés 250 autorisé 125 ans d'instruction et ses 742 éoliennes consomment déjà 174 hectares sur le département. Monsieur le rapporteur. de petite ampleur ou de grande ampleur. Si c'est une grande ampleur, ce sera nécessairement d'ampleur nationale et ayant vocation. Intégrer à notre compte. En tous cas une haute définition. En attendant donc défavorable sinon retrait. Monsieur le Ministre. Idem si les de petite ampleur il n'emporte pas de consommation d'artificialisation et si les de grande ampleur. Il rentre dans la catégorie telle que vient d'être défini, donc il est satisfait. C'est ça. Donc demande de retrait monsieur saumon. J'entends les réponses qui ont été donné à la fois par le rapporteur à la fois par le ministre et le ministre, il m'a pas répondu sur justement si vous savez que c'est les préfets qui délivrent les permis de construire. C'est donc bien l'État qui les, selon les les instructions qui lui sont données du ministère. Est-ce que vous allez donc faire l'économie aussi que vous demandez aux collectivités de réduire de moitié, là où il y a déjà énormément d'éoliennes si sur 20 15 ans, nous avons 700, 140 70 hectares. Est-ce que vous allez réduire la possibilité d'en avoir encore davantage ceux qui polluent les l'environnement et qui impacte. Grandement le département de la Somme en particulier. Ça n'est pas un sujet qui a directement à voir avec le zéro artificialisation nette pour la raison que je viens d'écrire, puisque la taille de l'éolienne emporte ou le fait qu'elle ne soit pas considéré comme de l'artificialisation si elle est trop petite, où le fait qu'elles ont dans les grands projets d'envergure nationale. Donc finalement vous m'interrogez, en lieu et place d'Agnès Pannier-Runacher et dans la continuité des débats qui ont eu lieu sur l'accélération des énergies renouvelables. Je suis persuadé qu'elle vous avez répondu à cette occasion sur un sujet qu'il connaît infiniment mieux que moi. Bien je vais donc soumettre aux voix l'amendement 154 rectifié bis avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient. Il n'est pas adopté le 36 rectifié Madame Berthet. On se présente, Monsieur le Ministre. Cet amendement. Oh ce que la nature des projets considérés d'ampleur nationale ou européenne et d'intérêt général majeure prévue au 7 de cet article soient précisées par un décret afin d'offrir une sécurité juridique suffisante aux porteurs de projet. Sur le rapporteur. Oui, monsieur le président. Chers collègues, c'est précisément. Ce que nous avons voulu éviter le pouvoir réglementaire. Et faire en sorte que pouvoir législatif le liquidateur ne peut pas ça pleinement sa sa sa fonction il apporte une la meilleure définition possible, c'est ce qui nous paraît être le cas à l'article IV. Donc ce sera un retrait sinon défavorable. Le. Monsieur le Ministre. Je suis assez favorable à cet amendement parce qu'il permettrait au contraire de revenir à l'article 181 que vous avez rejeté tout à l'heure et ça nous permettrait de fixer, par décret, ce qui avait dans l'amendement législatif mais donc je comprends la position du rapporteur mais favorable. Donc, avis favorable du gouvernement défaveur. Les la prévention. Ah je vais suivre l'avis du rapporteur, excusez-moi monsieur le Ministre, suit l'avis de mon collègue et retirer l'amendement. Donc, l'amendement est retiré. Nous passons à 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Monsieur Vial. Télé2. Oui. Merci monsieur le président je je vais présenter si vous voulez bien, donc les deux amendements le le 120 est un amendement de repli par rapport à l'amendement 119. j'ai dit tout à l'heure ce que je pensais des objectifs de de cette loi et et Dusan mais je pense avoir compris. Les les objectifs que que poursuivait la la la mission de la commission spéciale j'ai l'honneur de participer, c'est-à-dire de d'essayer de d'améliorer le texte actuel sans remettre en cause les les fondements principaux et en évitant le plus possible des dérogations qui rendrait. De difficile. La lecture, la lecture globale et l'atteinte des objectifs par ces amendements. J'ai souhaité justement répondre à cette à cette attente mais permettre également de prendre en compte les besoins. Incidence des projets d'intérêts nationaux parce que effectivement, Monsieur le Ministre, quand on décide un projet d'intérêt national, il y a des conséquences sur les territoires des impacts sur les territoires des conseils des dommages collatéraux de de de cette décision en terme de logement en terme d'infrastructures qui sont rendues nécessaires. Je prends un exemple, quand vous décidez de mettre en place une centrale nucléaire dans un territoire rural. Si vous avez 6000 employés sur cette centrale il va falloir les les personnes qui vont y travailler, créer un certain nombre d'infrastructures. Les amendements que qui sont proposés ici disent tout simplement que lorsqu'on décrète ou lorsqu'on décide d'un projet d'intérêt national, on étudie l'impact de ce projet sur le territoire et le cas échéant on peut permettre d'avoir une enveloppe complémentaire pour permettre de prendre en compte les incidences de ce projet pour, pour le rendre tout simplement réalisable, je dis bien le cas échéant puisque si on est en Île-de-France ou si on est sur un territoire rural la l'impact. Qui peut être pris par le territoire n'est pas forcément le même, donc on est sur. Sur un, un une enveloppe complémentaire qui permet de ses projets tout simplement efficient sur sur le territoire. Je je je profite juste Monsieur le Président pour expliquer la différence entre les 2 amendements. Le premier amendement. Permet de dire que les projets d'internationaux et cette enveloppe complémentaire sont pris sur le le le quota national donc ne ne compte pas dans le, le décompte de l'artificialisation des sols et l'amendement de repli permet de dire que le projet d'international et en dehors de l'enveloppe en revanche on impute sur l'enveloppe régionale donc mutualiser l'effort ni au niveau de la soleil sur la solidarité pardon régional ces ces efforts complémentaires qui seront nécessaires sur le territoire parce que effectivement ils auront aussi une traduction sur les territoires. Donc ça c'est un amendement de repli mais effectivement et le, le premier permet de de prendre en compte dans son ensemble le projet d'intérêt national, je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Avis de la commission. Monsieur le président. Et et, mes chers collègues, alors. Sur les deux amendements en effet alors je comprends parfaitement ce qui est exposé par notre collègue c'est Cédric Vial. J'avais un doute au départ sur l'enveloppe foncière complémentaires. Je persiste à avoir ce doute sur le fait de savoir si cette enveloppe complémentaire du fait de son impact pour réintégrer un grand projet et sortir potentiellement de comptes nationale maintient ce doute là. Et y compris sur sur sur l'amendement. En revanche, si ça peut faire l'objet d'une mutualisation régionale j'en comprends là l'intention.

Et réitère ici et. Indique. Toutefois qu'à titre personnel je vois un intérêt du fait des explications de notre collègue au deuxième un amendement donc ce sera un avis très personnel que c'est ce que ce sera le seul. Un doute Un doute pour Olivier Paccaud et l'inter-régionale IT c'est le deuxième doute. Positif. Que j'aurais ce soir moi je réitère très très défavorable. Ce que dit la Commission sur les deux amendements. Et en ce qui me concerne. Une sagesse favorable. Plein de nouveaux concepts ce soir sur le va. Monsieur le Ministre. Défavorable sur le 119 pour des raisons qui ont déjà été évoqués plutôt favorable sur le 120, à une limite. Près. Là on est dans l'article qui traite des grands projets d'envergure nationale et la catégorisation qui permettent d'aller délimiter des grands projets régionaux elle existe aussi dans le texte et ce qu'on a besoin d'un amendement qui prévoit une identification pour savoir si ça doit être rattaché à l'enveloppe régionale, alors que la liberté de de la collectivité régionale, ça peut être de conserver une enveloppe pour accueillir ce type de projets, sans qu'on ait besoin d'avoir un processus législatif qui rajoute des et donc dans l'esprit plusieurs interventions du sénateur via le ce soir sur pourquoi complexifié, ce qu'on pourrait rendent simple on donne de la souplesse. Je pense qu'il y a sans passer par cet amendement. La possibilité de le faire à une échelle régionale et que c'est même plutôt intelligent de garder une soupape pour identifier les projets pour les rattacher cette catégorie sans passer par l'objet d'un vote dans le corps du texte. merci. Est ce que vous maintenez les amendements monsieur Vial, allez-y. L'explication de vote. Mais, merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre, pour, pour ces explications, je pense en effet qu'on touche là à quelque chose de très sensible et et d'indispensable et très attendu sur les territoires parce que les gens les les élus sur le territoire ont peur des conséquences de ces projets qu'on qui pourraient se voir imposer et pourrait même. Aller contre certains projets ou considérer qu'il y aurait une double peine sur des projets qui leur seraient imposées et qui en plus viendrait empêcher tout développement endogène de leur territoire parce que les quelques cas passer de construction qu'ils ont, qu'ils auraient serait consacrée à autre chose que le développement qu'ils qu'ils auraient souhaité donc ces problèmes semblent me semble important. Jean j'entends ce que vous dites, Monsieur le Ministre. Mais il me semble justement que le fait de préciser même si c'est dans l'enveloppe régionale que ça fait partie du projet finalement et que quand on va déterminer l'enveloppe régionale et quand on va déterminer la manière dont on va les répartir. Il faut prendre en compte avec le projet les conséquences que ce projet peut avoir sur le territoire et vérifier ses capacités les capacités du territoire à pouvoir l'absorber ou à le développer. C'est pour ça que ça me semble important de le préciser jouera un amendement similaire tout à l'heure sur les projets d'intérêts régionaux. L'article 5 par cohérence voilà donc je me range. Suite aux discussions que nous venons d'avoir et elle est à la vie, notamment du rapporteur je je retire l'article 119 le l'amendement 119 pardon et je maintiens l'article 120 et je compte sur vous, mesdames et messieurs, chers collègues.

il est favorable à l'amendement 120 de. Du collègue Vial. Qui est contre.

149 présentée par. Notre collègue bonhomme je lui propose de présenter les trois dans la foulée. Merci, merci Monsieur Président oui le comme ça a été dit multiples fois la lutte contre l'artifice des sols et l'occasion. Importante de lutter contre l'étalement urbain et contre la dispersion des ménages de manière anarchique, Lausanne. De même, peut accélérer la politique d'aménagement durable du territoire de notre pays. Ainsi, en proposant de sortir du décompte quelques secteurs stratégiques sur lequel il est cohérente d'encourager l'émergence. Et une Et une dynamique de projets pourraient ainsi s'enclencher. Aussi il semblerait cohérent efficient dans ce cas d'exclure les périmètres des ORT dont l'objet même et de retrouver une dynamique locale pour des communes qui ont une vocation de centralité. Un engouement vertueux pour les OAT pourrait voir également le jour ça c'est le moment de 146 147 propose lui d'exclure les quartiers de de gare du décompte dans la mesure évidemment où l'un des objectifs Dusan et de lutter contre le réchauffement climatique en diminuant le CO2 et ainsi favoriser la voiture et le 249, lui propose d'exclure les périmètres des stations de transports publics comme le tramway ou encore les lignes régionales de bus. pardon avis du rapporteur sur ces trois amendements. Défavorable. Monsieur le président. Défavorable à vide. Monsieur le Ministre. Défavorable. Donc il y a un double avis défavorable sur ces trois amendements je vais soumettre aux voix. L'un après l'autre. Le 246 qui est pour.

En précisant qu'une liste et une enveloppe foncière nationale nécessaires à la réalisation de grands projets d'envergure nationale ou internationale sont définies en s'appuyant notamment sur des listes établies par les préfets de région, élaboré à partir des CPER de la politique immobilière de l'État et de ses plans prévisionnels pluriannuels d'investissement sont considérés comme projet d'envergure nationale. Tous les projets en maîtrise d'ouvrage de l'État directe ou délégués les projets menés par ces agences ou établissements publics une enveloppe du foncier consommée par ces grands projets, dans les 10 ans précédant la promulgation de la loi est établie et permet de piloter d'atteindre la trajectoire foncière et lutte contre l'artificialisation merci.

À partir essentiellement de la politique qu'il mène. Or ces projets peuvent rentrer. Selon moi, dans les critères prévus par le présent article ce sera défavorable. Avis défavorable de la commission. Monsieur le Ministre. Défavorable du gouvernement la maîtrise d'ouvrage par l'État n'est pas un indice suffisant, qu'il s'agit d'un grand projet d'envergure nationale et donc je redemande le retrait sinon le rejet, la liste est trop large.

Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Mes chers collègues. Nous avons examiné 89 amendements il aurait 135 examiner. Je vais lever la séance. La prochaine séance aura lieu mercredi 15 mars. À 15h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.